La séance est ouverte.

Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

à l'approche du rendez-vous référendaire, nous avons, vis-à-vis de nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie, mais aussi par respect pour ceux qui, dans leur diversité, ont scellé avec courage et lucidité les accords de Matignon-Oudinot, puis négocié et signé l'accord de Nouméa, l'ardente obligation de tout mettre en oeuvre pour que le résultat de cette consultation, terme du processus institutionnel qu'ils ont engagé, soit incontestable. Nous avons en effet vis-à-vis de cette génération d'hommes et de femmes- j'ai en particulier le souvenir d'un homme dans cet hémicycle -, qui, au-delà des blessures de l'Histoire, ont permis à la Nouvelle-Calédonie d'accomplir, dans le respect de leur diversité et des valeurs de la République,

L'unanimité rencontrée dans cet hémicycle lors de l'examen des articles montre, et je ne puis que m'en réjouir, la volonté de la Haute Assemblée de garantir cette légitimité, qui est la marque des principes que nous défendons ensemble et de l'attachement

manifestement pas s'y opposer ; il n'est pas logique d'être contre ... Cependant, je voudrais tout de même formuler un certain nombre de réserves, en particulier

de la démocratie, c'est : « Un homme, une voix. » C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme. Or on fait exactement le contraire ! Actuellement, des Français nés en France et habitant depuis plusieurs années en Nouvelle-Calédonie sont privés du droit de vote.

: en Corse, il y a des gens qui voudraient que les Français nés sur le continent ne puissent pas voter ! Veuillez conclure ! Ça, c'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je m'abstiendrai.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, prévue par l'accord de Nouméa de 1998, la mise en oeuvre de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie nécessite de transcrire dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le résultat de l'accord politique obtenu au sein du comité des signataires de l'accord de Nouméa, tenu le 2 novembre 2017. Le dépôt tardif du texte sur le bureau du Sénat a introduit une importante contrainte temporelle, avec laquelle nous devons composer compte tenu du nombre important de mesures réglementaires à publier et des délais de recours à respecter avant l'expiration du délai prévu par l'accord, au mois de novembre 2018. le Conseil d'État n'a pas manqué de souligner un calendrier particulièrement serré. Depuis 1998, les tensions se cristallisent essentiellement autour de la composition de la liste électorale spéciale rassemblant les électeurs habilités à prendre part à la consultation sur la pleine souveraineté, ses partisans dénonçant l'exclusion de près de 23 000 Kanaks sur 90 000 en âge de voter, soit une part non négligeable du corps électoral total, qui est de 160 000 personnes. C'est pourquoi nos collègues Gérard Poadja et Pierre Frogier, ainsi que les députés Philippe Gomès et Philippe Dunoyer, plaident auprès des partenaires politiques locaux et de l'État la nécessité de procéder à l'inscription d'office de ces quelque 11 000 natifs du pays sur les listes électorales. La conciliation entre une telle préoccupation et la nécessité de permettre aux nouveaux résidents français de prendre part à la vie démocratique explique la coexistence de trois listes électorales distinctes en Nouvelle-Calédonie. Conformément à la volonté exprimée lors du XVI comité des signataires de l'accord de Nouméa, le projet de loi organique soumis à notre examen comprend diverses mesures pour garantir la légitimité du scrutin et favoriser la plus large participation des « populations intéressées » à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, assurant ainsi la sincérité de la consultation à venir. Le projet de loi organique traduit fidèlement la volonté commune des signataires de l'accord de Nouméa, des représentants des institutions calédoniennes et des formations politiques locales. La commission des lois a approuvé ce texte, moyennant quelques améliorations, auxquelles le groupe du RDSE a souscrit en commission. Lors de l'examen du texte la semaine dernière, j'ai défendu deux amendements émanant du président du groupe du RDSE, Jean-Claude Requier. Le premier visait l'information des électeurs que nous considérions comme nécessaire sur les modalités d'exercice du droit d'option,

de voir précisé le vote par procuration. Je rappellerai que l'avis du Conseil d'État souligne une fois encore les lacunes de l'étude d'impact fournie par le Gouvernement s'agissant des mesures relatives au régime des procurations. L'objectif de notre groupe était d'attirer l'attention de tous les acteurs sur la question des procurations. Mme la ministre de l'outre-mer, que je tiens à remercier, nous a apporté les éléments nécessaires pour nous rassurer sur les modalités pratiques d'information. C'est donc en toute logique que nous avons décidé de retirer ces deux amendements. Sur le plan strictement législatif, le projet de loi organique entre dans le cadre en vigueur. Pourtant, notre groupe attire l'attention du Gouvernement sur l'organisation même de la consultation. Le président de la commission des lois, dont j'ai salué l'engagement dans ce dossier, s'est rendu personnellement en Nouvelle-Calédonie au début du mois de janvier, pour s'assurer que le dispositif prévu correspondait bien à la volonté de toutes les forces en présence. en présence. Il a souligné en commission des lois, le 7 février dernier, que cette consultation comportait des risques pour la concorde civile en Nouvelle-Calédonie. Notre collègue Gérard Poadja indiquait également qu'une consultation mal préparée pourrait provoquer des tensions ethniques et politiques. Ainsi, en contribuant à rendre le résultat incontestable, les dispositions de ce projet de loi organique sont de nature à favoriser une consultation référendaire apaisée. Toutefois, j'aimerais y ajouter une autre préconisation, qui concerne le texte même de la question posée. Notre groupe insiste sur l'impérieuse nécessité que la question posée pour la Nouvelle-Calédonie soit claire et sans ambiguïté. Les seules réponses possibles doivent être le « oui » ou le « non La formulation de la question ne doit pas être l'occasion d'ouvrir un autre débat. Sinon, les efforts déployés pour rendre incontestable cette consultation voleraient en éclat, et nous risquerions d'ouvrir une crise politique majeure, que ce territoire n'a pas le luxe de s'offrir aujourd'hui. j'ai noté la semaine dernière votre détermination à faire en sorte que cette question posée soit d'une « indispensable clarté », pour reprendre vos propos. Le groupe du RDSE salue cette prise de position du Gouvernement. ne nous y trompons pas : cette consultation ne réglera pas le sujet institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci ne se résume pas à savoir si le territoire doit ou non devenir un État souverain. La réalité est beaucoup plus complexe. Au-delà de l'aspect strictement législatif et institutionnel, j'aimerais insister sur le fait que tout doit être fait pour que cette consultation ne crée pas une fracture au sein de la population. En réalité, ce qui se joue depuis quelques décennies en Nouvelle-Calédonie, c'est un « mieux vivre ensemble », que j'associe au troisième pilier de notre devise républicaine : la fraternité. Dans un contexte que nos collègues calédoniens ont très bien décrit, cette consultation risque de créer une nouvelle fracture entre des populations qui cherchent une nouvelle voie pour mieux vivre ensemble. Au-delà de la loi, se joue là le destin de populations qui souhaitent avant tout trouver un juste équilibre dans le respect de leurs réalités respectives. Nous ne prétendons pas avoir la solution. Je crois que, sur ce sujet, il appartient aux Calédoniens eux-mêmes de construire cette troisième voie du « mieux vivre ensemble ». Celle-ci ne passe pas seulement par la loi. Mes chers collègues, vous aurez remarqué que nous avons parlé de « population calédonienne », et non de « peuple calédonien Cette dernière notion renvoie du point de vue constitutionnel à une souveraineté qui n'existe pas encore à cette heure. C'est ce que le rapporteur Philippe Bas a précisé à la fin de nos échanges la semaine dernière en se plaçant sur plan strictement juridique. Il n'y a donc aujourd'hui ni souveraineté actée ni, par conséquent, peuple calédonien. Nous ne saurions qu'inviter les responsables politiques à ne pas entretenir de doute sur ce sujet en employant parfois des termes juridiques inappropriés.

aussi déterminant que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de la France, tout est affaire de point de vue ; et d'abord, cher Philippe Bas, de point de vue législatif. Oui, résolument, nous allons voter ce texte, bien préparé par son rapporteur, qui s'est déplacé en Nouvelle-Calédonie. Nous le voterons parce qu'il est la traduction législative et juridique d'un compromis politique sur le corps électoral. Il donnera une force incontestable au résultat référendaire dans quelques mois. Toutefois, mes chers collègues, nous ne pouvons pas nous contenter de ce point de vue juridique, législatif. Il faut absolument que nous relevions l'horizon, que nous passions du point de vue juridique à un point de vue politique. En effet, dans cette affaire si déterminante, la question n'est pas seulement celle de la légitimité d'une consultation référendaire. référendaire. C'est celle, finalement beaucoup plus importante, d'un accord fondamental ; c'est celle du devenir de la Nouvelle-Calédonie et de la France ; c'est celle d'une association

le seul dont on ne connaît pas le point de vue, le seul qui refuse obstinément de s'engager, c'est l'État ; c'est le Gouvernement ! Vous avez déclaré voilà quelques jours que l'État devait être un partenaire et un acteur de la discussion. Très bien

on peut parfaitement respecter la neutralité d'un point de vue technique, électoral, tout en exprimant du fond du coeur politiquement l'attachement que nous avons, que vous devez avoir pour la Nouvelle-Calédonie

pas seulement constitutionnelle, mais républicaine, née des propos du Premier ministre sur le sol calédonien ! Quand le Premier ministre dit qu'il y a un « peuple calédonien » amené à s'exprimer « souverainement cela signifie qu'il existerait un peuple calédonien distinct du peuple français ! Mais au nom de quoi ? Au nom de quelle réalité ? Parce que la Nouvelle-Calédonie se trouve aux antipodes ? Parce qu'une partie de la population a la peau sans doute un peu plus foncée que la nôtre en métropole ? Non, bien sûr ! C'est ignorer ce qu'est la France. La France, c'est cet effort multiséculaire pour conjuguer ce qu'il y a de particulier dans chaque homme

Le troisième risque est celui de la distanciation. N'ajoutons pas à la distance géographique avec la Nouvelle-Calédonie une autre distance, plus grave celle-ci : une distance civique. Au fond,

dans la France en Nouvelle-Calédonie ni dans la Nouvelle-Calédonie dans la France ; nous voulons et nous croyons dans une nouvelle Calédonie française ! Nous y croyons au

peut intégrer dans son destin toutes les petites patries charnelles pour composer la grande patrie française ! La parole est

l'organisation de ce référendum est un engagement de l'État. Dans notre démocratie,

C'est une raison supplémentaire de souligner que l'organisation de ce référendum est un moment très important. La décision appartient et appartiendra aux Calédoniens, et personne d'autre ne peut décider de l'avenir de leur territoire. étant, à titre personnel, je souhaite que la Nouvelle-Calédonie continue à enrichir le paysage des outre-mer français

C'est finalement au sein de la République française que nous avons cette formidable occasion de soutenir notre cause, celle des territoires d'outre-mer. Ce n'est pas facile tous les jours

La France a cette formidable chance d'être d'ores et déjà présente dans tous les bassins océaniques, sur tous les continents, quand d'autres puissances

que nous pourrons continuer à défendre la cause des outre-mer dans la France !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte pour lequel nous nous apprêtons à voter est très important. À l'évidence, il va recueillir l'assentiment de notre assemblée. Cependant, revenons sur le sujet de ce projet de loi organique. Il s'agit aujourd'hui non pas de modifier le corps électoral pour le futur référendum en Nouvelle-Calédonie, dont la composition répond à des critères fixés en 1998, mais bien de traiter de la question de l'inscription d'office d'électeurs pour participer au scrutin, afin que celui-ci comptabilise un maximum d'électeurs potentiels. Je ne reviendrai pas ici sur l'ensemble des remarques et des mises en garde que j'ai formulées la semaine dernière ; je me limiterai simplement à quelques observations sur les modifications apportées par notre chambre haute.

Aussi, au sujet des dispositions ajoutées à ce texte par le Sénat, je m'interroge tout de même sur l'intention, semble-t-il tacite, de la disposition prévue à l'article 3 , qui, « dans le but d'éviter les dysfonctionnements liés à l'usage très répandu du vote par procuration tend à encadrer le recours à cette modalité de vote lors de la consultation d'autodétermination. Quels sont les dysfonctionnements visés ? visés ? Il aurait été intéressant de les étayer. En effet, cela nous laisse une impression désagréable de tromperie- mais de qui et pourquoi ? Quoi qu'il en soit, les justificatifs nécessaires qui seront requis pour participer au scrutin par procuration et qui seront définis par décret en Conseil d'État après consultation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ne devront pas nuire à la participation la plus large de la population sur place. Certes, des bureaux de vote seront délocalisés à Nouméa pour faciliter le droit de vote des habitants des communes insulaires, mais aucune sorte de « contrepartie » n'aurait dû être exigée. Mes chers collègues, vous conviendrez qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties que le taux de participation à ce scrutin soit le plus élevé possible, pour une issue la plus démocratique qui soit. Aussi, ce genre de disposition visant à complexifier le droit de procuration aurait-il pu être évité. En ce sens, nous serons attentifs au décret d'application. Ma seconde remarque porte sur le décret en Conseil des ministres qui fixera le texte de la question posée aux électrices et aux électeurs lors de la consultation. Nous nous félicitons de l'amendement adopté visant à consulter le Congrès de Nouvelle-Calédonie sur le décret en question. Nous porterons donc une attention toute particulière à la teneur de la question qui sera posée. nous savons bien, mes chers collègues, que dans ce genre de consultation chaque mot revêt son importance. Il s'agira, là encore, d'être le plus objectif possible et de retranscrire l'esprit de l'accord de Nouméa, porteur de paix entre les parties représentées. Il devra en être de même quant aux règles propres à la campagne audiovisuelle qui régiront le temps d'antenne de chacun, et plus largement sur les conditions dans lesquelles va se dérouler la campagne électorale. Il est en effet essentiel qu'elle soit en phase avec la législation existante, mais la plus équitable, la plus citoyenne et la plus démocratique possible. Encore une fois, je le répète, l'équilibre entre indépendantistes et loyalistes, bien que consolidé par trois décennies de paix, reste fragile de plus d'un siècle d'histoire douloureuse. Quelle que soit l'issue du scrutin, et nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir dans cet hémicycle, l'État français aura la responsabilité et le devoir d'accompagner les Calédoniennes et les Calédoniens, dans leur diversité, vers le choix d'avenir d'avenir qu'ils auront fait. Pour l'heure, gageons que l'organisation de cette consultation sera une réussite, en apportant avec notre vote unanime notre pierre à l'édifice de ce long processus institutionnel. La parole

ayant déjà eu l'occasion de m'exprimer longuement en commission et lors de la discussion générale sur le projet de loi organique qui nous est aujourd'hui soumis, je rappellerai simplement l'esprit et la lettre d'un texte fondateur pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France, dans ses relations avec notre pays : le préambule de l'accord de Nouméa. Un préambule qui éclaire le texte que nous examinons aujourd'hui. On a su, au travers de ce préambule, mettre des mots sur les non-dits de notre histoire commune. On a su parler des « ombres et lumières » de la période coloniale pour reprendre la belle formule de l'accord. On a su reconnaître que le peuple kanak, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie était un peuple colonisé, qui avait été marginalisé aux frontières géographiques, économiques et politiques de son propre pays, selon le texte de l'accord. Un peuple dont l'identité a été niée dans ses fondements mêmes : ses langues, son lien à la terre, son rapport au temps et au monde. C'est pourquoi cette reconnaissance du fait colonial était indispensable. une autre reconnaissance l'était tout autant : celle des populations qui, tout au long de la période coloniale, venues d'Asie, d'Océanie et d'Europe dans le cadre de la colonisation libre ou pénale, ont, au fil du temps, dans des conditions particulièrement difficiles, mis en valeur la Nouvelle-Calédonie et contribué à son développement. Ces populations ont, là aussi, par leur participation à la construction du pays, acquis une légitimité à vivre en Nouvelle-Calédonie et à décider de son avenir. Le texte que nous allons adopter aujourd'hui est la traduction politique et juridique du préambule de l'accord de Nouméa. Il apporte une définition ultime au corps électoral référendaire qui devra se prononcer dans quelques mois sur l'avenir de notre pays. Ce texte contribue à la définition d'un peuple, le peuple calédonien, ce peuple de toutes les couleurs et de toutes les cultures, qui, par les hasards de l'histoire du monde, est en train de se construire dans une petite île du Pacifique en Mélanésie. Un peuple qui a appris à conjuguer populations autochtones et populations venues d'ailleurs. Comme l'a souligné dans une belle formule le président du Sénat, notre collègue Gérard Larcher, lors de sa venue devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 23 février 2016

et s'incarne dans la citoyenneté inscrite dans la loi organique du 19 mars 1999. » Oui, monsieur le président du Sénat, vous avez vu juste : malgré les difficultés, « l'unité du peuple calédonien » a toujours prévalu. Et je souhaite de tout mon coeur que, malgré les inévitables tensions, il en soit de même au lendemain du référendum, pour que les Calédoniens puissent continuer à construire leur destin commun, dans la France et dans la paix. Mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce projet de loi organique. La parole est à M.

Nous sommes amenés aujourd'hui à faire un travail législatif avec une grande modestie, car ce travail est issu

La décolonisation est aujourd'hui le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Les communautés qui vivent sur le territoire ont acquis, par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie, une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement.

L'équilibre a été trouvé. Il fallait permettre aux électeurs des îles Loyauté de venir voter à Nouméa. Pour la première fois, des communes vont organiser sur le territoire d'une autre commune des bureaux de vote pour leurs ressortissants

dans le rapport de Sophie Joissains, de Jean-Pierre Sueur et de Catherine Tasca. Cet esprit a aussi permis des acquis importants sur la culture et la coutume kanake, un pouvoir très fortement décentralisé, une organisation très spécifique. Mes chers collègues, ce référendum est une étape, mais il pourra être suivi, le cas échéant, si un tiers du Congrès de Nouvelle-Calédonie le demande, de deux autres référendums dans les deux années consécutives. C'est selon moi à ce

faudra faire des propositions, notamment organisationnelles, s'inspirant de ce qui est en place aujourd'hui- c'est fondamental. Cela permettra sans doute aussi d'éviter les deux autres référendums, s'ils sont demandés

Cette forme politique, dit-il, est « manifeste en Nouvelle-Calédonie ». Il ajoute : « Je pense en particulier à la nécessité des contrepoids et des équilibres entre les institutions Cette force politique, cette capacité d'équilibre, de contrepoids entre les institutions, doit aussi fonder notre République. Si elle a permis depuis trente ans la paix en Nouvelle-Calédonie, j'espère, madame la ministre, que le Premier ministre saura s'en souvenir dans les réflexions actuelles sur la révision constitutionnelle : il faut préserver l'équilibre entre les institutions et l'existence de contrepoids

celui des modalités de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. La route a été longue et semée d'embûches. ans après les accords de Matignon, vingt ans après les accords de Nouméa, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie nourrit encore de nombreuses interrogations, parfois même des tensions. Depuis des années, la question du corps électoral de cette consultation perturbe le débat public. Les citoyens français vivant aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit l'origine de leur présence sur le sol calédonien, doivent pouvoir, dans des conditions indiscutables, participer à la consultation. C'est ce que prévoit le texte soumis à notre approbation en ouvrant le plus largement possible le corps électoral et en répondant aux particularismes géographiques de certaines communes. Lors de la séance, à l'écoute de nouvelles propositions, le Gouvernement a proposé l'adoption de deux amendements inscrits dans le prolongement de ces mesures un premier point concerne le remboursement des dépenses de campagne, pour assurer la transparence et la régularité des scrutins ; un second point concerne la répartition des temps d'antenne et d'intervention pendant la campagne, de manière qu'une stricte équité entre toutes les parties soit respectée, sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Lorsque ce texte nous a été présenté, la semaine passée, les deux orateurs de notre groupe ont souligné le travail d'apaisement du Gouvernement, ce que l'on pourrait appeler la « méthode Philippe », très largement saluée. Notre collègue Jérôme Bignon, membre du groupe de contact sur la Nouvelle-Calédonie créé sur l'initiative du président Gérard Larcher, a voulu saluer tout particulièrement le travail accompli par les acteurs locaux, notamment par nos collègues parlementaires calédoniens du Sénat et de l'Assemblée nationale. Notre collègue Jean-Louis Lagourgue, quant à lui, a souhaité rappeler l'équilibre fragile récemment établi. Il convient de penser dès à présent à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, quel que soit le résultat de cette consultation, afin que le dialogue puisse se poursuivre entre toutes les parties, dans un climat serein. Penser l'avenir, c'est d'abord trouver ce qui unit la population calédonienne. Le sénateur Pierre Frogier, acteur historique de ces débats, a plusieurs fois évoqué l'éventualité de la tenue de « palabres à l'océanienne sortes d'états généraux de l'avenir calédonien, rassemblant l'ensemble des forces politiques et la population locale. Le Gouvernement a montré sa disponibilité et sa responsabilité dans ce dossier, en prêtant l'oreille aux revendications de l'ensemble des acteurs du processus, en dépit de la grande complexité des sujets. Penser l'avenir, c'est ensuite continuer de prévoir : prévoir l'avenir économique, industriel et social de la Nouvelle-Calédonie. Plusieurs fois, la question de l'industrie du nickel a été évoquée dans ces débats. Il est donc nécessaire qu'une feuille de route soit rapidement dressée, ainsi que le comité des signataires l'a souligné au mois de novembre 2017. Ce projet de loi, mes chers collègues, c'est la première pierre de la fondation sur laquelle bâtir la Nouvelle-Calédonie de demain. Une grande partie de la jeunesse en Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui en proie à des difficultés d'emploi et de santé. Il faut envisager des mesures sérieuses d'accompagnement. Tout est à construire : une école plus inclusive, donnant sa chance à chacun ; une société plus tolérante et moins sujette aux addictions et aux violences ; une diminution de la criminalité ; enfin, une hausse de l'emploi.

et soyons respectueux de leur choix, car l'avenir heureux ne peut se bâtir que dans le respect mutuel des uns et des autres.

démocratique et transparente, appuyée sur un corps électoral respecté où chacun trouve sa place et peut s'exprimer. Madame Madame la ministre, mes chers collègues, il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, au scrutin public solennel

Jacky Deromedi, Guy-Dominique Kennel et Victorin Lurel, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Je rappelle qu'une seule délégation de vote est admise par sénateur. Je déclare le scrutin ouvert

au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie,

Le Sénat a adopté le projet de loi organique

des affaires européennes. Je souhaite évoquer la crise migratoire à laquelle doit faire face l'Europe, et notamment la France. C'est un sujet de préoccupation majeur qui cristallise les passions et les peurs. Dans plusieurs États européens, les questions de l'identité et du contrôle des frontières redeviennent centrales et font l'objet de toutes les instrumentalisations. Attisé par la crise migratoire, l'euroscepticisme gagne partout du terrain et pas seulement en Europe centrale et orientale, ce qui, de mon point de vue, n'est pas une bonne chose. Nous connaissons les conditions de l'accord avec la Turquie, qui a certes sclérosé les flux de Méditerranée orientale, mais d'autres voies d'arrivée demeurent. Et ils sont encore des centaines de milliers de migrants, notamment en Libye, vivant dans des conditions inhumaines, livrés aux trafiquants. Le Président Macron qui, durant sa campagne, pour des raisons électorales, avait donné des gages à son camp sur les questions migratoires semble opérer aujourd'hui un retour au réalisme en souhaitant- enfin -clairement distinguer le cas des demandeurs d'asile de celui des migrants économiques. Pourtant, lors d'une récente rencontre à Bruxelles, j'ai entendu des officiels de haut niveau de la Commission m'expliquer que, face à un phénomène historique auquel l'Union européenne ne pouvait se soustraire et, par ailleurs, totalement bénéfique pour combler pour combler une natalité européenne en berne, il était impératif de se montrer souples et d'accueillir le plus grand nombre. Dès lors, que pèsera la position française face à cette vision irresponsable qui semble se dessiner à Bruxelles ?

nous nous apercevons qu'en l'espace d'un an- l'année 2017 -, les flux migratoires ont diminué de moitié.

La ligne est claire : être capables d'accueillir celles et ceux qui peuvent bénéficier de l'asile parce qu'ils sont victimes de persécutions dans leur territoire, dans leur pays, pour des raisons ethniques, religieuses ou politiques, et

de la désintégration sociale. Entre inefficacité et angélisme, il me semble que l'Union européenne met elle-même en place les conditions d'une défiance à son égard, dont je crains qu'elle ne soit difficile à arrêter. C'est regrettable.

Emmanuel Macron s'est engagé à réformer l'assurance chômage, promettant la mise en place d'une indemnisation universelle pour les démissionnaires et les indépendants. Nous attendons les conclusions des négociations entre les partenaires sociaux et le Gouvernement, et nous discuterons ensuite du projet de loi. Je m'inquiète, madame la ministre, de la prise en compte de la situation particulière des agriculteurs dans l'élaboration de vos futures réformes. Chaque semaine, plus de 200 exploitations disparaissent en France. Que deviennent les agriculteurs contraints d'abandonner leur activité ? Ils sont la plupart du temps démunis et sans perspectives. La semaine prochaine, toute la France agricole sera réunie à Paris. Cette France doute, madame la ministre. Son activité est remise en cause par les conséquences des traités CETA et MERCOSUR, par le reclassement des zones défavorisées simples, par les crises sanitaires à répétition et par la préparation de l'après-PAC 2020. Le rôle de l'État est de protéger les hommes et les femmes qui exercent ce métier difficile et ô combien essentiel. Qu'en est-il lorsque, malgré tous leurs efforts, ils doivent se résigner à abandonner une exploitation souvent familiale depuis plusieurs générations ? Il faut les accompagner, leur permettre de se reconvertir, leur redonner de l'espoir. Vous défendez les évolutions économiques et les mutations professionnelles. Vous devez aussi protéger les agriculteurs. Madame la ministre, comment comptez-vous répondre à cette urgence sociale ? Comment la situation des agriculteurs sera-t-elle prise en compte dans vos futures réformes ? La parole

Le Président de la République s'est engagé, en application de son programme, à ouvrir le bénéfice de l'assurance chômage aux travailleurs indépendants, ce qui inclut donc les agriculteurs. L'objectif est de protéger ceux qui s'engagent de façon entrepreneuriale dans une activité non salariée. Une chose est sûre : nous n'augmenterons pas les cotisations des travailleurs indépendants puisqu'ils contribuent désormais au régime d'assurance chômage à travers la contribution sociale généralisée, la CSG. Dans cette perspective, j'attends les propositions des partenaires sociaux, qui sont en cours de négociation. Sur ce sujet, l'État a bien sûr l'intention d'agir

Monsieur le Premier ministre, les Guyanais, en rébellion permanente contre un système qu'ils jugent inopérant dans les domaines les plus essentiels, notamment ceux de la santé, de l'éducation, de la sécurité et du développement économique, sont très préoccupés, voire « remontés » contre le rythme et l'état d'avancement des accords de Guyane, obtenus après deux mois de mobilisation d'une grande ampleur, une véritable révolution. Ils attendaient de la concrétisation de ces accords, signés par votre prédécesseur et confirmés par le Président Macron, des avancées notables, rapides dans certains domaines les plus vitaux tels la santé et la sécurité, puisque faisant partie d'un plan d'urgence. Certes, monsieur le Premier ministre, des mesures ont été prises dans le cadre de ces accords. Deux comités de suivi se sont même tenus, dont le dernier en septembre 2017, un mois avant la venue du Président de la République en Guyane. Mais depuis, certains critiques de l'action gouvernementale disent que les accords marquent le pas, tout semblant être suspendu aux assises des outre-mer, dont le calendrier de réalisation serait à plus longue échéance que celle qu'escomptaient les Guyanais. Cela est d'autant plus vrai que dans le même temps se tiennent les états généraux de Guyane. Tout cela crée une réelle confusion qui vient s'ajouter au sentiment d'exaspération, au « ras-le-bol », au fameux « », comme on l'exprime si bien dans notre langue guyanaise. Alors, manifestations, débrayages, grèves, violences urbaines et scolaires ont repris de plus belle et renvoient actuellement à la situation qui a précédé les événements de l'an dernier, ce qui fait craindre le pire. Aussi, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous apporter aux Guyanais des assurances sur le respect par votre gouvernement des accords de Guyane, et ce dans leur totalité, c'est-à-dire des garanties sur la prise en compte, à la fois, du plan d'urgence, du plan complémentaire et du projet institutionnel ou statutaire pour lequel ils opteront ? La parole

du Gouvernement pour la Guyane et, plus globalement, pour les outre-mer. Cette « page nouvelle de la relation entre la République et les outre-mer »-je cite ses mots -est celle de la responsabilité partagée.

dans ses responsabilités les plus fondamentales : la santé, la sécurité et l'éducation. Je sais aussi les aspirations de la population de Guyane à un modèle de développement plus équilibré.

J'en veux pour preuve la mobilisation exceptionnelle des crédits de l'État pour les constructions scolaires, notamment dans l'ouest guyanais : 250 millions d'euros engagés sur cinq ans pour les lycées et les collèges, et 150 millions d'euros sur dix ans pour les écoles. Nous allons redonner à la collectivité territoriale de Guyane de la capacité à investir pour l'avenir en recentralisant, conformément aux engagements pris par le Président de la République, les dépenses de RSA pour la Guyane. Dès 2017, dans le cadre du fonds d'urgence prévu par l'État, nous avons apporté 50 millions d'euros supplémentaires pour faire face à l'augmentation rapide, massive, de la dépense en Guyane. Nous allons évidemment poursuivre sur ce chemin. Mais la politique de l'État, monsieur le sénateur, vous l'avez dit et je pense qu'il est essentiel de l'avoir à l'esprit, ne se résume pas au plan d'urgence du premier trimestre 2017. Celui-ci a permis de répondre rapidement à l'urgence- c'est le cas de le dire ! -, quand l'avenir exige une construction de long terme. D'abord, un mot sur le pouvoir d'achat : dans beaucoup de collectivités d'outre-mer, le niveau de la taxe d'habitation est très élevé- c'est le cas en Guyane. Cette année, une grande partie des habitants des communes de Guyane pourront constater la baisse massive de cette taxe, compensée aux communes. Notre engagement en matière de sécurité est renforcé : la Guyane figure parmi les vingt départements reconnus comme prioritaires dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. En matière d'immigration- une question importante -, dans le cadre d'une expérimentation circonscrite à la Guyane, nous allons essayer, expérimenter, à compter de juin prochain, la réduction des délais d'instruction des demandes d'asile. Monsieur le sénateur, vous le constatez, nous avançons, nous agissons. Il est vrai, j'en conviens volontiers, qu'avant de nous engager très en avant et très loin, nous prenons le temps de la réflexion.

Ils le seront encore davantage avec le Livre bleu outre-mer qui marquera la conclusion des assises en mai prochain. Mme la ministre des outre-mer y est évidemment particulièrement investie.

ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et concerne la filière bois. Monsieur le ministre, notre pays est couvert de 16 millions d'hectares de forêt, soit 29 % du territoire. La France est à la tête de la troisième plus grande surface forestière d'Europe.

Or force est de constater que la filière a perdu depuis 15 ans 20 % de sa valeur ajoutée et 100 000 emplois. Elle pâtit d'un déficit commercial d'environ 6 milliards d'euros par an. L'augmentation des exportations, notamment vers la Chine, de bois brut non transformé pose la question de l'approvisionnement de la filière. En effet, de nombreuses scieries françaises sont contraintes de fonctionner en deçà de leur capacité. On constate qu'un certain nombre de pays forestiers concurrents ont contraint la fuite de cette ressource brute, donc non transformée.

Il est nécessaire, d'une part, de mettre en place une véritable politique volontariste et, d'autre part, d'assurer la cohérence des politiques publiques pour faciliter la valorisation locale du bois. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes sensible à cette problématique, pouvez-vous nous informer sur les mesures que vous entendez mettre en oeuvre pour répondre à ces défis et sortir la filière bois de la crise qui la ronge ?

dont je sais combien il est important pour chacune et chacun d'entre vous ici. Vous interrogez le ministre de l'agriculture sur un enjeu majeur, celui de l'avenir de la filière bois et de la gestion plus globale de la forêt, avec tous les emplois que vous évoquez. Effectivement, nous savons que, outre l'enjeu d'aménagement du territoire que représente la gestion forestière, il y a aussi ces 440 000 emplois. Vous avez raison, la Fédération nationale du bois s'inquiète aujourd'hui de l'exploitation massive de grumes. Ce n'est pas un phénomène nouveau : vous l'avez souligné, il a commencé voilà une dizaine d'années. Vous avez aussi mentionné les engagements qui avaient déjà été pris, sous l'autorité de Stéphane Le Foll, par le gouvernement précédent pour que l'on puisse avoir les moyens de défendre cette économie essentielle pour notre territoire. d'un durcissement des conditions administratives et sanitaires liées à l'export de grumes, avec, par exemple, l'augmentation du tarif de la certification sanitaire par les services de l'État ou l'interdiction des produits phytosanitaires dangereux, afin qu'il y ait une juste concurrence entre les bois de nos producteurs et ceux qui sont importés. Je citerai aussi, comme vous l'avez fait, le label de l'Union européenne utilisé par l'Office national des forêts, l'ONF, qui doit garantir l'origine des grumes dans les pays de l'Union européenne. concerne les mesures que nous devons mettre en oeuvre, c'est par exemple l'élargissement de ce label UE à l'ensemble de la forêt privée, qui, aujourd'hui, n'est pas dans ce cadre. Nous souhaitons, dans les semaines qui viennent, faire en sorte que cela puisse se mettre en oeuvre, et mettre en place une adhésion des producteurs à des coopératives forestières. Nous voulons également contribuer à améliorer le dialogue dans la filière. L'ONF a été chargé a été chargé de la mise en oeuvre de ces outils par Stéphane Travert, qui conduira, dans les prochains mois, un travail pour que ceux-ci soient renforcés dans le cadre du Grand plan d'investissement.

abandon des lignes non rentables, soit 9 000 kilomètres de rail ; filialisation du fret ; privatisation des trois établissements constituant la SNCF ; ouverture à la concurrence totalement libre pour le TGV ; abandon du statut des cheminots, et j'en passe. Madame la ministre, vous l'avez dit, le n'est pas une option, le rail doit se moderniser et se développer par l'investissement. Il a besoin de financements nouveaux, d'une vision renforcée de ses missions au service de l'aménagement du territoire et du droit à la mobilité pour répondre aux besoins croissants de la population et des nouveaux modes de vie et de déplacement. À l'inverse, ce rapport sonne comme une insulte à nos territoires ruraux, périurbains, car supprimer des lignes régionales, c'est détruire la cohésion et l'égalité territoriale. La décision de fermeture de lignes par l'État est une ineptie, tout comme le transfert sur les compétences régionales : les collectivités déjà asphyxiées ne pourront assumer des axes de transports essentiels et structurants pour nos concitoyens. Avec la parution de ce rapport, la « start-up Nation » érigée comme modèle d'avenir par votre gouvernement montre ses limites ou plutôt ses priorités : libéralisme décomplexé face à la solidarité des territoires, ou encore aménagement européen face à l'aménagement national. La création de déserts ferroviaires va encourager les gens à utiliser le transport routier, alors que l'argument écologique est avancé. Votre gouvernement souhaitait faire des transports du quotidien sa priorité absolue. Qu'il commence par ne pas abandonner les transports en région, en évitant la création d'un service public à deux vitesses ! Ma question sera simple comptez-vous reprendre les préconisations de ce rapport qui condamne le service public ferroviaire et met au ban de nombreux habitants, considérés dès lors comme des Français de seconde zone ?

notre service public ferroviaire joue clairement un rôle essentiel, avec plus de 11 000 trains qui circulent chaque jour et plus de 4 millions de voyageurs. Mais force est de constater que ce service public rencontre de graves difficultés, avec une qualité de service qui n'est pas au niveau attendu par les Français, avec des coûts qui ne cessent de croître, avec une dette qui augmente de 3 milliards d'euros par an. Pourtant, nous n'avons jamais consacré autant d'argent au service public ferroviaire, 20 % de plus aujourd'hui qu'il y a dix ans. Pourtant, je connais l'engagement des cheminots, dans leur mission de service public, au service des voyageurs. Pourtant, tous nos concitoyens sont attachés au service public ferroviaire. C'est face à cette impasse, à ces contradictions, que le Gouvernement a souhaité disposer d'un rapport posant une vision globale sur le secteur public ferroviaire. Ce rapport pose un constat sévère, mais malheureusement juste, ... Juste ? On pourrait en discuter ! ... sur les difficultés que rencontre notre système ferroviaire. Aujourd'hui, les propositions sont sur la table et, avec le Premier ministre, nous avons engagé une concertation avec tous les acteurs. À l'issue de ces concertations, nous annoncerons la méthode et le calendrier. S'agissant des petites lignes- ce terme n'est pas adapté, car je sais que ce sont des lignes essentielles pour beaucoup de nos concitoyens -, je le dis clairement : nous avons prévu d'investir 1,5 milliard d'euros dans les contrats de plan. Ces engagements ne seront pas remis en cause. Ce n'est pas à Paris que se décidera l'avenir de ces lignes, mais dans les territoires, avec les régions, au plus près des besoins des voyageurs ! La parole

Durant cette attente, je songeais à une révolution positive des transports, dans la continuité des propos du Premier ministre qui évoquait « une véritable refondation de la SNCF Je songeais au maillage territorial pour tous du XIX siècle qui aurait été transcendé et adapté aux défis du XXIsiècle et des nouvelles mobilités. Je songeais à une véritable cure de jouvence pour notre SNCF, ce pilier de notre République, qui a contribué à unifier le territoire. Mais nous en sommes loin ! Il y a bien sûr quelques bonnes idées et bons principes, mais, pour l'essentiel, nous sommes dans les vieilles recettes, et dans un conformisme libéral qui a montré ses limites appliquées au service public. Qu'avez-vous est la transformation en société anonyme de l'EPIC SNCF Réseau et Mobilités, au motif d'un endettement trop important, qui n'a évidemment pas été provoqué par les cheminots mais bien par les choix d'investissement de l'État. société anonyme, le statut des cheminots ne pourra être amené à évoluer que par la négociation, et non par des effets d'annonce. Madame la ministre, à la suite de ce rapport, dans lequel la place de l'usager n'est encore que trop peu prise en compte, je vous pose plusieurs questions au nom du respect de la parole donnée. Souhaitez-vous maintenir cette approche française de la structuration du territoire par les mobilités ? Pouvez-vous confirmer que les haltes TGV existantes ne seront pas supprimées alors même que certaines ont été cofinancées par les collectivités territoriales, comme dans ma région Grand Est ? Enfin, quels moyens seront dégagés pour financer les investissements pour les fameuses lignes à faible trafic prévus dans les contrats de plan État-région ? Quels types de financements peut-on imaginer afin de donner un avenir à ces lignes Mme la ministre chargée des transports. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jacquin, je voudrais vous redire que l'engagement du Gouvernement, c'est bien d'améliorer la mobilité pour tous les Français, dans tous les territoires. Les assises nationales de la mobilité ont, à cet égard, permis de faire remonter de très nombreuses propositions, y compris la nécessité de sortir des zones blanches de la mobilité. Vous savez sans doute que 80 % de notre territoire n'est pas couvert par une autorité organisatrice de la mobilité mobilité : par conséquent, personne ne s'occupe de proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle dans ces territoires. C'est vrai ! Le service public ferroviaire a clairement un rôle important à jouer dans notre politique de mobilité au service de tous les territoires. Mais, comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes face à des impasses, à des coûts qui ne cessent de croître, à une dette qui ne cesse d'augmenter et à une qualité de service qui ne répond pas aux attentes de nos concitoyens. Nos concitoyens le savent bien : ceux qui vivent avec angoisse le fait de prendre un train et qui se demandent s'ils vont arriver à l'heure au travail ; ceux qui constatent que, pendant qu'on inaugure quatre lignes à grande vitesse au cours des dix-huit derniers mois,

auquel nous allons consacrer 36 milliards d'euros dans les dix prochaines années, soit 10 millions d'euros par jour pendant dix ans, de refonder le modèle ferroviaire que le Gouvernement a souhaité ce rapport pour définir une stratégie globale en termes de service public ferroviaire. La parole

au nom d'un impératif environnemental, que l'on peut partager, mais qui a entraîné une montée des prix à la pompe et du chauffage. Je suis élu d'un territoire rural et je tiens à vous alerter sur les difficultés rencontrées par les habitants, les professionnels du transport et les agriculteurs. Les habitants des zones rurales ont besoin de leur véhicule pour se rendre à leur travail et ont souvent de nombreux kilomètres à faire, quelquefois une Nombre d'entre eux possèdent des véhicules diesel, puisque les gouvernements précédents incitaient à acheter ces voitures, et n'ont pas les moyens financiers d'en changer. Par ailleurs, les véhicules électriques aujourd'hui adaptés aux territoires ruraux, en raison d'un manque d'accès à des bornes et d'un coût trop onéreux. Pour défendre activement la ruralité, fragile, il faut conserver le niveau du pouvoir d'achat dans ces territoires. La hausse du prix du gazole ne permet pas aux salariés de profiter des avantages financiers liés à la suppression

vous avez raison, les transports sont trop souvent vécus comme une injustice entre citoyens et entre territoires. C'est la raison pour laquelle notre politique de mobilité doit répondre à cette réalité, et permettre de lutter contre les fractures territoriales et l'assignation à résidence. C'est bien pour cela que dans la loi d'orientation des mobilités, que nous présenterons prochainement au Parlement, il sera notamment proposé d'assurer la couverture complète de notre territoire par des autorités organisatrices de la mobilité, d'offrir des solutions alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle, de soutenir la mobilité inclusive et de développer les plateformes de conseil en mobilité. Dans ce même objectif de lutte contre les fractures territoriales, les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures prévoient un plan de désenclavement du territoire pour sortir des promesses, reportées de contrat de plan en contrat de plan, de mise à niveau de notre réseau routier. S'agissant de la transition énergétique, notre ambition est bien qu'elle profite à tous nos concitoyens. Le développement de l'autonomie des véhicules électriques permet d'élargir leur domaine de pertinence. Aujourd'hui, 22 000 bornes de recharge ouvertes au public ont été déployées dans tout le territoire. Nous accompagnons

de cette année, une aide de 1 000 à 2 000 euros, pour l'achat de véhicules Crit'air 1 ou 2. C'est bien pour accompagner la mobilité de tous nos concitoyens et pour prendre en compte les exigences du transport routier que nous avons proposé dans la loi de finances pour 2018 des mesures d'aide et de soutien au suramortissement pour les véhicules GNV et le gel de la TICPE pour le GNV de nos transporteurs routiers. La parole

le Gouvernement sur trois sujets importants qui concernent l'avenir de la viticulture, pilier de notre patrimoine culturel. Tout d'abord, la transmission des exploitations. La viticulture est frappée par la hausse du prix du foncier et l'arrivée d'investisseurs extérieurs. La profession propose qu'un repreneur soit exonéré de droits de mutation sur l'outil d'exploitation, dans l'objectif de préserver un tissu d'entreprises familiales dans nos vignobles. Ensuite, la création d'une réserve de gestion des risques. Le mécanisme existant de la déduction pour aléas n'ayant jamais remporté l'adhésion des agriculteurs en raison notamment de sa complexité, la profession demande la mise en place d'un dispositif visant à permettre aux entreprises de se constituer une « réserve d'autofinancement » avec des mesures fiscales adaptées. Enfin, l'engagement des exploitations viticoles dans la certification environnementale. Les vignerons sont de plus en plus nombreux à intégrer dans leurs pratiques une meilleure prise en compte de l'environnement. Or le coût d'une certification est très lourd pour les petites exploitations. Afin d'encourager et d'accompagner les viticulteurs il conviendrait de leur accorder un crédit d'impôt. Monsieur le Premier ministre, entendez-vous intégrer les présentes attentes de la profession viticole dans le projet de loi de Avant de conclure, je souhaite rebondir sur un précédent débat. Les représentants de la filière vitivinicole que j'ai récemment rencontrés se veulent des acteurs des politiques de prévention et de pédagogie de nos produits et revendiquent un devoir de responsabilité. Je considère qu'ils sont donc totalement légitimes à être associés avec les pouvoirs publics sur les stratégies nationales de la santé qui les concernent. Je vous remercie de prendre en considération cette demande.

projet de loi de finances pour 2018 est apparue la nécessité d'une réflexion globale sur la fiscalité agricole. Le ministre de l'économie et des finances ainsi que le ministre de l'agriculture ont pris l'engagement de mener une concertation de l'ensemble des acteurs du secteur, en associant étroitement les parlementaires. Vendredi dernier a eu lieu le lancement de cette mission de concertation en présence des représentants des organisations syndicales et professionnelles agricoles. Le groupe de travail, que nous avons voulu transpartisan, comprend dix députés et dix sénateurs, désignés selon la représentation et la représentativité des groupes devant chaque assemblée et au choix des deux assemblées. Sur ce sujet, comme sur d'autres, il nous paraît possible et souhaitable de s'affranchir des clivages politiques. L'objectif est d'aboutir à des propositions ambitieuses et cohérentes qui trouveront leur place dans le prochain projet de loi de finances. Les enjeux de cette réforme visent notamment à répondre aux points que vous avez soulevés concernant les préoccupations des viticulteurs : il s'agit, en particulier, d'améliorer la résilience des entreprises en encourageant la gestion des risques et des aléas par la constitution de provisions ou d'épargne de précaution de renforcer la compétitivité des entreprises agricoles en favorisant les systèmes de production plus performants ; de favoriser la transmission des entreprises agricoles, sujet que vous avez mentionné ; enfin, de prendre en compte la diversification des activités agricoles.

Monsieur le ministre, le site de Vallourec à Tarbes est dans une situation critique : en décembre dernier, le groupe Vallourec, dont le principal actionnaire n'est autre que l'État, annonçait la vente des sites à une entreprise américaine. Vous le savez, deux sites ne sont pas concernés par cette reprise, Cosne-sur-Loire, sur lequel ma collègue sénatrice de la Nièvre, Nadia Sollogoub, vous a déjà interpellé, et le site de Tarbes, pour lequel Viviane Artigalas, que j'associe ici à ma démarche, et moi-même sommes mobilisées. Les délais imposés par Vallourec pour une reprise des sites concernés fixent la date butoir au 28 février prochain : sans candidat sérieux déclaré, l'entreprise fermera, laissant plus de 50 salariés sans emploi sur le site de Tarbes. Les Hautes-Pyrénées ont payé le prix fort de la désindustrialisation : 7 000 emplois industriels ont été sacrifiés en trente ans au profit de la métropole toulousaine, qui attire à elle toutes les activités. Vallourec est, au-delà d'un bouleversement humain et social, un symbole : celui de l'abandon d'une stratégie industrielle française. Il est temps que l'État intervienne pour endiguer la désertification industrielle des territoires ruraux, où la qualité de vie et le savoir-faire technique sont pourtant au rendez-vous. Le 26 janvier dernier, le délégué interministériel aux restructurations venait à notre rencontre pour nous assurer que des projets de reprise étaient à l'étude. À huit jours de l'échéance fixée par le groupe Vallourec, nous n'avons toujours aucune assurance d'une reprise : je vous laisse imaginer la détresse des salariés face à cette situation. Nous pouvons pourtant aujourd'hui compter sur un outil de production adapté ; un client, Nexter, dont l'importance pour l'armée française est plus que stratégique, qui assure 36 % de la production du site ; enfin, un véritable savoir-faire du personnel, ouvert à une diversification de l'activité. Aussi, monsieur le ministre, l'État consentira-t-il enfin à faire pression sur le groupe Vallourec en sa qualité d'actionnaire pour qu'il ne fasse pas tomber le couperet du 28 février sur la tête des salariés, et permette ainsi à un repreneur de bâtir un projet industriel sérieux dans un délai raisonnable ?

d'une partie des sites, mais pas de ceux de Cosne-sur-Loire et Tarbes, qui n'ont pas été repris par National Oilwell Varco, le repreneur du reste de l'activité. Comme vous l'avez dit, dit, Jean-Pierre Floris, délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, s'est déplacé à Tarbes le 26 janvier dernier pour visiter le site et rencontrer les salariés. Il a également reçu le directeur général de la société Vallourec Drilling le 16 février dernier pour faire le point sur la recherche de repreneurs. Je peux vous assurer que des moyens importants sont mis en oeuvre par la société avec un cabinet spécialisé pour donner, d'ici à la fin du mois de février, la visibilité aux salariés quant à l'avenir du site de Tarbes. Des contacts entre la société et des repreneurs potentiels sont en cours. Deux d'entre eux ont visité le site ces derniers jours. Vallourec travaille avec les repreneurs potentiels en vue d'aboutir rapidement au dépôt d'offres de reprise indicatives qui ouvriraient la voie à des discussions approfondies sur ces projets. Je vous assure que le Gouvernement et les services de l'État maintiennent leur pleine vigilance afin de permettre la poursuite d'activités sur ce site.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. La politique agricole commune est l'un des fondements de la politique européenne. L'idée, portée depuis 1957, est simple. Les pays dotés d'un potentiel agricole important bénéficient de transferts nets de la part des pays européens qui ne peuvent subvenir à leurs besoins alimentaires. Il s'agit d'une mesure de solidarité, d'une mesure juste. Il convenait de le rappeler. Au cours de ces dernières décennies, malgré les coups de boutoir répétés de certains pays non agricoles et des hautes autorités bruxelloises pour en finir avec la PAC, la France a toujours résisté. La défense des agriculteurs en Europe a toujours été une ligne rouge infranchissable. Il semble pourtant que le Président de la République et votre gouvernement se préparent, pour la première fois dans l'histoire, à rompre avec cette fermeté et à accepter une baisse du budget de la PAC.

le moment de cet abandon serait vraiment bien mal choisi, car nos agriculteurs sont au bord de l'asphyxie- le département du Lot-et-Garonne, dont je suis issue, connaît aussi, hélas, ce désastre. Baisser le budget de la PAC de 10 %, de 15 % voire de 30 %, comme le proposent certains, constituerait une véritable trahison des agriculteurs français. Monsieur le ministre, une baisse du budget de la PAC est-elle envisagée ? Si oui, le Président de la République sera-t-il alors le premier Président français à l'accepter ? Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat, personne au Gouvernement ni- j'en suis convaincu -au sein de la Haute Assemblée ne souhaite abandonner la PAC.

la PAC est et restera l'une de nos priorités. La France porte évidemment une vision ambitieuse de cette politique intégrée, qui est aussi, je vous le rappelle, la première politique européenne défendre une PAC ambitieuse, responsable, qui protège nos agriculteurs et qui libère nos entreprises agricoles, pour transformer le système de production. En effet, il ne suffit pas d'avoir une approche quantitative, il faut également avoir une exigence qualitative sur ce sujet. Ce n'est la France devra être offensive pour maintenir le budget de la politique agricole commune, indépendamment de l'impact du Brexit. Il faudra aussi obtenir une simplification de sa mise en oeuvre pour les

de sommes d'argent, il faut aussi profiter de cette PAC pour que celle-ci soit porteuse d'une ambition environnementale renforcée, permettant la rémunération des services environnementaux. Vous n'aimez pas l'environnement ? ? Je suis assez surpris que vous n'admettiez pas le rôle majeur du monde agricole en matière de préservation de l'environnement ; or il faut bien évidemment rémunérer l'engagement de nos agriculteurs à ce sujet. Aussi, je vous le dis, la France portera cette ambition, cette exigence financière,

socialiste et républicain. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale. Imaginez, un seul instant, que vous deviez, après une vilaine chute, marcher avec des béquilles pendant quatre mois. Heureusement, on aurait inventé de nouvelles béquilles plus adaptées, qui vous permettraient de bien mieux vous déplacer, mais, voilà, à cause de leur coût, on ne pourrait vous les donner que pendant le premier mois.

Ce dédoublement des cours préparatoires constitue une belle ambition, mais à condition d'y mettre les moyens. Il n'est pas raisonnable de penser que les classes rurales soient une variable d'ajustement pour récupérer des postes ; il n'est pas raisonnable de liquider le dispositif plus de maîtres que de classes » sans laisser le temps nécessaire à son évaluation ; il n'est pas non plus raisonnable de puiser dans les effectifs de remplacement. Monsieur le ministre, le résultat de votre politique oppose les territoires entre eux, alors qu'il faut tenir compte de la spécificité de chacun. Très bien ! Par exemple, dans le département dont je suis élu, la Somme, vous envisagez de supprimer une classe dans la commune de Fressenneville ou encore dans celle d'Eaucourt-sur-Somme.

des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, n'imaginons pas, regardons la réalité plutôt que le fantasme, et n'alimentons pas le fantasme sur un sujet aussi important que l'éducation de nos enfants.

Concrètement, cela signifie que, partout en France, dans la ruralité, y compris dans votre département, il y aura davantage de professeurs par élève. Nous n'aurons donc pas fait le choix de soutenir les élèves les plus fragiles dans les quartiers les plus difficiles contre la ruralité ; ces chiffres-là sont faux.

15 nouveaux postes de professeur. Dans ce département, le vôtre, la carte prévisionnelle, telle qu'elle a été présentée par les services de l'inspection d'académie, prévoit 38 fermetures de classe- vous avez raison, il y aura des fermetures de classe -, contre

aveugle et muet pour considérer que, quand il y a des baisses d'effectif, il faut maintenir des classes ; je crois que personne ne peut tenir ce discours-là. Par conséquent, nous voyons bien qu'il est inopportun et injuste d'opposer la ruralité aux quartiers, notamment dans votre département, monsieur le sénateur,

ma question concerne les fermetures de classe unique en zone rurale, plus précisément à Havange, en Moselle. Cette commune a une classe unique à tous les cours avec dix-neuf élèves. Au motif d'une légère baisse à la rentrée, l'Éducation nationale vient de programmer sa fermeture. Ainsi, dans la ruralité, on exige dix-neuf élèves pour maintenir une classe unique à tous les cours, alors que, dans les quartiers urbains dits « sensibles », le Gouvernement a fixé le seuil à douze élèves pour des classes à un seul cours. C'est donc clair, monsieur le ministre : on déshabille les zones rurales au profit des quartiers à problèmes ! Oh ! Monsieur le ministre, pourquoi refusez-vous que, dans la ruralité,

des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, depuis des années, il y a un décalage entre le nombre d'élèves dans les classes rurales et le nombre d'élèves dans les classes urbaines, et c'est une bonne chose. Je suis moi-même élu des Alpes-de-Haute-Provence, j'étais confronté à cette réalité, celle de la distance, de la difficulté de l'accès à l'école. Je pense que, depuis des années, jamais un urbain n'a prétendu qu'il fallait contester cette réalité, qui avantage, en nombre d'élèves par classe par rapport au professeur, le monde rural ; mais vous êtes en train de faire la mécanique inverse.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur du débat disposera d'un temps de parole de dix minutes, y compris la réplique, puis le Gouvernement répondra pour une durée équivalente.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est un honneur d'introduire ce débat sur les conclusions du rapport de la délégation aux droits des femmes relatif à la situation des agricultrices, un sujet méconnu, alors même que 30 % des exploitations sont aujourd'hui dirigées par des femmes, que 36 % des salariés agricoles sont des femmes, et que, depuis toujours, les femmes apportent un tribut essentiel à l'agriculture. Notre rapport est issu d'un travail de longue haleine, accompli entre février et juillet 2017. Il a été porté par une équipe de six corapporteurs représentant le Sénat dans sa diversité politique de l'époque ; notre délégation est en effet attachée à la méthode du consensus. Ce rapport donne largement la parole au terrain, au travers du témoignage de plus de cent agricultrices, rencontrées à l'occasion d'un colloque organisé au Sénat, il y a tout juste un an, le 22 février 2017, puis dans le cadre d'auditions et de tables rondes, ainsi qu'au cours de quatre déplacements en en Vendée, en Bretagne, en Haute-Garonne et dans la Drôme. Le rapport analyse la situation des agricultrices dans sa globalité, au travers de toutes les étapes de leur parcours professionnel formation, installation, statut, protection sociale, santé, engagement dans les organisations professionnelles agricoles, accès aux responsabilités et retraites. Il évoque aussi les difficultés spécifiques liées à l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale pour des femmes qui exercent un métier où la charge de travail est considérable et dont les contraintes d'organisation peuvent être aggravées par un accès parfois inégal aux services publics, aux soins et aux moyens de communication. Les constats du rapport rendent compte des échos que nous avons recueillis sur le terrain. Certains de ces ressentis concernent tant les femmes que les hommes et reflètent le malaise d'une profession que nous ne pouvions passer sous silence. Je souligne d'ailleurs qu'une résolution du Parlement européen sur les femmes et sur leur rôle dans les zones rurales, adoptée en mars 2017, rejoint les constats que nous avons établis dans notre rapport. Premier constat de la délégation : l'insuffisance des revenus et l'impression d'une dégradation régulière de la situation, tant pour les femmes que pour les hommes.

Autre constat : « Le métier a besoin d'être défendu », car il pâtit d'une image négative qui contribue à l'isolement du monde agricole. Christiane Lambert déclare encore : « Nous sommes la profession oubliée » En ce qui concerne les difficultés spécifiques aux agricultrices, il est important de rappeler que celles-ci sont les héritières d'une longue invisibilité. Le fait qu'elles aient longtemps été considérées comme « sans profession » nous a tout particulièrement interpellés. Par ailleurs, la crise oblige de nombreuses agricultrices à travailler à l'extérieur de l'exploitation pour rapporter un revenu, ce qui multiplie par deux leur charge de travail. Nous avons également voulu insister sur les obstacles que rencontrent souvent les jeunes agricultrices pendant leur parcours de formation et d'installation, qu'il s'agisse de l'accès aux stages, plus compliqué, semble-t-il, pour les jeunes filles élèves de l'enseignement agricole, ou de l'accès au foncier. Enfin, plusieurs points sont souvent revenus dans les témoignages reçus en lien avec l'isolement du monde rural : le besoin de solutions d'accueil des jeunes enfants et les conséquences très préjudiciables, particulièrement pour les femmes, de la désertification médicale. J'en viens maintenant à la présentation de nos 40 recommandations, adoptées à l'unanimité. visent notamment à adapter les critères d'attribution des aides à l'installation au profil atypique des agricultrices, qui exploitent des surfaces généralement plus petites que les hommes et s'installent plus tardivement qu'eux. Nous formulons également des propositions pour faire en sorte que les agricultrices bénéficient d'une retraite et d'un revenu décents c'est un prérequis de toute amélioration de la condition agricole. Ce point n'a même pas fait débat entre nous ; il s'agit là d'une question de dignité. De la même manière, plusieurs de nos recommandations portent sur le statut des agricultrices, notamment sur le recensement des agricultrices sans statut- elles sont aujourd'hui entre 5 000 et 6 000 sur la sensibilisation du monde agricole au préjudice lié à l'absence de couverture sociale. En outre, nous avons été surpris de constater qu'à peine 58 % des agricultrices recourent au service de remplacement en cas de maternité. Cette proportion relativement faible s'explique soit par le coût du service de remplacement, soit par le fait que le profil du remplaçant ne correspond pas toujours aux attentes. Plusieurs de nos recommandations portent donc sur un meilleur accès au congé maternité pour les agricultrices, y compris en cas de grossesse pathologique. À cet égard, je me félicite du chantier ouvert par le Gouvernement pour harmoniser le droit à congé maternité selon les professions, ce qui devrait être, je l'espère, bénéfique pour les agricultrices. De façon plus générale, nous recommandons d'améliorer la communication sur les services de remplacement, et de sensibiliser les agricultrices aux bénéfices que peuvent leur apporter ces services, car ils leur sont indispensables, que ce soit pour les congés maternité, pour suivre des stages de formation continue ou pour l'exercice de mandats syndicaux ou dans les chambres d'agriculture. Enfin, un pan entier de nos recommandations concerne la nécessité de renforcer la reconnaissance des agricultrices, afin qu'émergent des modèles auxquels les jeunes filles- les agricultrices de demain -peuvent s'identifier. La mise à l'honneur des agricultrices peut passer par des remises de prix ou de trophées, comme l'a illustré notre colloque du 22 février 2017. Nous recommandons ainsi la poursuite et la généralisation à toutes à toutes les régions des « prix des femmes en agriculture ». Dans certains territoires, ces prix ont été abandonnés au moment de la réforme des régions : ils doivent être réactivés. Les remises de prix pourraient, par exemple, se tenir le 15 octobre, à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale ou, plus classiquement, le 8 mars. Je souhaiterais connaître le sentiment de la secrétaire d'État sur cette proposition, dont la mise en oeuvre, en lien avec les préfectures, ne me paraît pas hors de portée. En outre, nous avons pu constater le rôle décisif des réseaux d'agricultrices, tel le groupe Égalité-parité : Agriculture au féminin, de la chambre d'agriculture de Bretagne, en tant qu'élément essentiel de l'autonomie professionnelle des femmes, de la diffusion des bonnes pratiques et de prise de confiance en soi. C'est pourquoi l'une de nos recommandations vise à encourager la diffusion de tels réseaux dans d'autres territoires. Je conclurai par la question centrale de la place des femmes dans la gouvernance agricole. Si la proportion de femmes dans les chambres d'agriculture est en moyenne de 27 % sous l'effet de la loi du 4 août 2014, on constate que les bureaux de ces instances- qui, eux, n'ont fait l'objet d'aucune contrainte législative -demeurent très masculins. Nous proposons donc que la proportion d'un tiers de femmes, prévue par la loi du 4 août 2014, s'étende aux présidences de commissions et aux bureaux des chambres d'agriculture, comme aux instances dirigeantes des syndicats agricoles. Voilà, monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, une présentation sans doute trop rapide de notre rapport que je vous invite à lire en détail, ainsi que les actes de notre colloque qui a, voilà un an, rencontré un vrai succès. Je souhaite souligner que ce travail collectif a été très bien perçu et relayé dans les territoires et qu'il a suscité beaucoup de satisfaction, mais aussi d'attentes, de la part de nos interlocutrices. Toutefois, des recommandations n'ont de sens que si elles sont suivies d'effet.

nous avons eu l'occasion de le présenter au salon international des productions animales, le SPACE, de Rennes, en septembre 2017 avec quelques collègues, puis devant la commission nationale des agricultrices de la FNSEA, en décembre je voudrais relever que la prochaine session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, qui se tiendra dans quelques jours à New York, aura pour thème

Je me réjouis donc que, grâce à l'Union interparlementaire, je puisse participer à cette session et montrer l'intérêt que porte le Sénat français au thème central de cette réunion, dédiée aux femmes rurales. Très bien ! La parole est à Mme la secrétaire

Je salue l'esprit de consensus qui a guidé votre réflexion commune. Ce rapport est le fruit des échanges très constructifs que vous avez eus avec les agricultrices, les organisations professionnelles, les institutions sociales et les services de l'État. Je voudrais souligner la richesse du travail accompli, mais aussi l'importance des enjeux que nous aurons à relever collectivement pour faire progresser très concrètement l'égalité entre les femmes et les hommes partout en France, et particulièrement dans les territoires ruraux. Traditionnellement, le monde agricole a longtemps été considéré comme un milieu d'hommes en raison de la pénibilité physique des travaux, du temps de travail conséquent, des risques professionnels importants. Cette culture du risque fait partie de ce que l'Institut Catalyst appelle les « normes masculines du pouvoir bien plus valorisées dès l'enfance chez les petits garçons que chez les petites filles. La persistance de ces stéréotypes nous conduit à penser que la direction d'une exploitation, ou même seulement un investissement identique, à parts égales, des femmes dans tous les travaux agricoles ne peut- théoriquement -pas constituer une option pour elles. Et pourtant, comme votre rapport le montre parfaitement, les femmes occupent depuis longtemps une place de premier plan dans la vie des exploitations. C'est vrai ! Elles assument une part importante de l'emploi agricole et contribuent, de manière privilégiée,

Garantir aux femmes les mêmes droits que ceux des hommes dans le secteur agricole constitue donc un enjeu fondamental pour notre pays. Comme vous le savez peut-être, je suis originaire de Corse et élue de la Sarthe. Je sais donc à quel point les agricultrices sont essentielles à la vie et au dynamisme de la France.

cette égalité en acte lors de ma visite du domaine agricole de Valle, premier GAEC de Corse géré par un couple à parité. Plus récemment, lors du voyage officiel du Président de la République en Corse, de nouveau,

La haute fonctionnaire en charge de l'égalité au ministère de l'agriculture a activement participé à vos travaux. À la demande du ministre, elle a travaillé en étroite collaboration avec le service des droits des femmes et de l'égalité pour que cette feuille de route 2018-2020 intègre l'essentiel des propositions présentées dans ce rapport. Je pense tout particulièrement au soutien renforcé aux projets portés par les femmes, à la promotion de la parité dans les instances représentatives, ou encore à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu rural. Le ministre de l'agriculture et moi-même assurerons, évidemment dans la durée, la mise en oeuvre et le suivi de cette feuille de route. Conformément à vos recommandations, cet enjeu d'égalité est pleinement pris en compte au sein de l'enseignement agricole qui développe une pédagogie innovante sur les sujets liés à l'égalité filles-garçons. aurons-nous l'occasion d'y revenir au cours de nos échanges. Comme vous le savez, le Président de la République a choisi de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. L'annonce faite le 25 novembre dernier à l'Élysée est la traduction d'un engagement pris par le Président durant sa campagne, lorsqu'il déclarait : « La loi a changé ; maintenant c'est la vie des femmes qui doit changer ». Pour ce faire, il faut agir au plus précis, au plus concret des situations de chaque territoire. L'objectif est le même partout et pour tous : l'égalité entre les femmes et les hommes, ni discutable ni négociable. Toutefois, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif peuvent différer d'un territoire à l'autre, en fonction de plusieurs paramètres l'accessibilité des services publics, la richesse du tissu associatif, la situation économique et sociale, les particularités géographiques. Repenser la manière dont le service public s'organise partout en France, au plus près des réalités des territoires, voilà l'un des enjeux.

L'objectif de ce Tour de France est d'identifier précisément les besoins, les attentes des femmes, pour adapter les politiques publiques à la diversité des situations, mais aussi pour partager les bonnes pratiques et faire connaître les dispositifs innovants qui existent à l'échelle des territoires. six mois, près de 850 ateliers ont été organisés dans toute la France- métropole et outre-mer -et ont rassemblé plus de 55 000 personnes. À l'issue de ces échanges, je constate que les préoccupations et les demandes qui se sont exprimées dans les zones rurales rejoignent de nombreuses recommandations formulées dans votre rapport, notamment en matière de droits sociaux. Au cours des deux dernières décennies, la protection sociale des femmes exerçant une activité agricole s'est améliorée, en particulier avec la fin du statut de conjointe participant aux travaux

telle réforme permettrait de compléter l'évolution vers l'égalité des droits, avec la limitation progressive des statuts secondaires et du statut des aides familiaux.

Vous suggérez, dans votre rapport, de limiter à cinq ans la durée du statut de conjoint collaborateur. Cette piste de réflexion doit être étudiée à condition qu'elle corresponde aux attentes des agricultrices. Les femmes qui, aujourd'hui encore, travaillent sur une exploitation sans aucun statut doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Mon collègue ministre de l'agriculture et moi-même serons aussi particulièrement vigilants à garantir les droits des femmes agricultrices à certaines périodes charnières de leur vie. L'arrivée d'un enfant fait partie de ces moments particuliers, votre rapport le souligne. La réglementation permet aujourd'hui de se faire remplacer pour une durée égale

Je sais les agricultrices très attachées aux dispositifs existants. Je ne doute pas que cette mission saura être attentive à la recherche d'un équilibre entre ce qui existe et ce que nous pouvons proposer pour améliorer la protection de ces femmes quand elles deviennent mères. autre moment particulier de la vie des femmes. Le plan de revalorisation des petites retraites agricoles, avec l'attribution de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire, a surtout bénéficié aux femmes, ce qui est une bonne chose. Toutefois, malgré les efforts consentis, il faut reconnaître que les retraites agricoles sont plus faibles que celles des autres régimes, notamment pour les agricultrices. Autant de constats qui illustrent la pertinence de votre recommandation visant à limiter l'accès au statut de collaboratrice. Je vous confirme que cette question sera portée par le ministère de l'agriculture à la faveur des travaux sur la réforme globale des retraites. évidemment, les agricultrices aujourd'hui en activité bénéficieront des évolutions qui seront retenues dans le cadre de cette réforme. C'est la raison pour laquelle, dès la semaine prochaine, je lance, dans la Vienne, notamment avec Jean-Paul Delevoye, une réflexion sur la retraite des femmes.

à la question de la place des femmes et de leurs conditions de vie dans les zones rurales. La parole

d'État. Ce rapport est le début d'un long travail. Le Sénat et la délégation aux droits des femmes resteront vigilants pour suivre l'application de ces mesures. Très

moyenne, à 1 300 euros par mois, contre 800 euros pour les agriculteurs et 500 euros pour les agricultrices, quand le minimum vieillesse est de 900 euros par mois, pour un travail à temps plein.

à celles des chefs d'exploitation. Le montant des retraites allouées aux conjoints d'exploitants a été au coeur des dispositifs de revalorisation des retraites agricoles. Depuis 2011, les collaboratrices d'exploitation sont affiliées au régime de retraite complémentaire obligatoire, le RCO, ce qui contribue à à améliorer légèrement le niveau de retraite de ces femmes jusqu'alors affiliées au seul régime de base. Les femmes sont les principales bénéficiaires du plan de rattrapage des retraites agricoles qui s'est concrétisé dans la loi du 20 janvier 2014. Depuis 2014, 66 points gratuits de RCO sont attribués aux conjoints et aux aidants familiaux justifiant d'une durée minimale d'assurance au titre des années antérieures à la création du régime, et ce dans la limite de dix-sept années. Le montant de la retraite des chefs d'exploitation ayant effectué une carrière complète a été porté à 75 % du SMIC net par la création d'un complément différentiel de RCO mis en oeuvre au 1 janvier 2015. S'agissant de l'action du Gouvernement, sachez que, ce matin même, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire chargé de la réforme des retraites, a réuni un groupe de travail sur la réforme des retraites,

madame la présidente de la délégation, chère Annick, mes chers collègues, elles s'appellent Karen, Catherine, Jacqueline, Émeline, Marie-Blandine, Élodie, Sarah, Nathalie, Ghislaine, Brigitte, Perrine, Marie-Christine, Anne, Sylvie Elles vivent dans les départements du Lot, du Doubs, du Maine-et-Loire, du Gers, de Loire-Atlantique, de Haute-Garonne, de la Drôme, des Ardennes, d'Ille-et-Vilaine, du Rhône, de Haute-Marne, du Morbihan, du Loiret, de Meurthe-et-Moselle, de Vendée. Elles ont en commun d'être « femmes en agriculture ». Elles élèvent des ovins, des vaches laitières et allaitantes, des lapins, des porcs, des chevaux, des volailles. Elles produisent des céréales, des légumes, des fruits, du vin. Elles sont engagées, parfois militantes, dans les organisations professionnelles agricoles, présidentes de lycée agricole, présidentes de chambre d'agriculture, présidentes de section féminine, élues municipales, départementales, régionales, et ancienne sénatrice, pour l'une d'entre elles. Elles, ce sont les femmes que j'ai eu la chance de rencontrer, parmi d'autres, en tant que corapporteur, aux côtés de mes cinq collègues, à l'occasion du colloque organisé ici même ou lors de nos déplacements. Elles ont fait de leur passion un métier choisi et assumé. Elles se caractérisent par leur esprit d'ouverture. Elles ont le souci de la recherche de valeur ajoutée, une sensibilité aux questions environnementales et sociétales. Certaines accueillent des touristes ou pratiquent la vente directe. Elles sont vives d'esprit et épanouies. Pourtant, ce rapport met en exergue les conditions parfois difficiles dans lesquelles elles vivent leur activité, de la formation à la retraite, à l'instar de leurs homologues masculins sur certains aspects. nous avons l'obligation collective de faire vivre ce rapport et ses quarante recommandations pour reconnaître les carences et insuffisances, pour redonner du sens à ce noble métier et de l'espérance à celles qui l'ont choisi. Il nous appartient désormais, législateur, ministre de l'agriculture- pour l'enseignement agricole -, chambres consulaires, mutualité sociale agricole, banques, coopératives agricoles, collectivités locales et autres acteurs de l'agriculture et de la ruralité de tout mettre en oeuvre pour obtenir des résultats à la hauteur des espoirs suscités.

Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la mise en oeuvre des recommandations du rapport d'information établi par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Les services du ministère de l'agriculture ont vocation à examiner très concrètement, une par une, les suites qui peuvent être réservées à l'ensemble des recommandations À la demande de Stéphane Travert, la haute fonctionnaire en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère de l'agriculture, qui a participé activement à vos travaux en 2017, a élaboré une feuille de route sur l'égalité des droits 2018-2020 qui intègre l'essentiel de vos recommandations dont elle s'est inspirée pour faire ses propositions : soutien renforcé aux projets portés par les femmes, promotion de la parité dans les instances représentatives décisionnelles, formation et accompagnement des jeunes filles vers les métiers de l'agriculture, lutte contre les violences faites aux femmes en zone rurale. L'ensemble du ministère en assurera la mise en oeuvre et le suivi concret dans la durée. J'ajoute que ces enjeux sont pleinement pris en compte au sein de l'enseignement agricole qui développe depuis peu une pédagogie innovante sur les sujets liés à l'égalité entre filles et Par ailleurs, certaines des recommandations émises dans ce rapport avaient déjà fait l'objet de réflexions ayant conduit à inscrire des dispositions spécifiques dans les textes au cours des dernières années- loi retraite de 2014, loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ...

Marche. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la délégation, mes chers collègues, femme d'agriculteur éleveur dans le Morvan, conjointe collaboratrice depuis la loi de juillet 1999 instituant ce statut, mère de trois enfants, je me sens particulièrement concernée par ce débat. Comme toute femme, une agricultrice doit pouvoir s'épanouir dans sa vie professionnelle et familiale. Le domaine le plus clivant entre hommes et femmes est celui de la maternité. D'où mes différentes Comment les pouvoirs publics peuvent-ils mettre en place un service de remplacement entièrement pris en charge permettant à ces agricultrices d'avoir une grossesse sereine sans risque de complications, de soigner leur enfant quand il est malade ? Comment allez-vous permettre le développement de solutions d'accueil pour la petite enfance en milieu rural ? Quelles structures innovantes, prenant en compte les contraintes des métiers de l'agriculture, ce qui implique de pouvoir recourir à des formules souples-

cette équité entre, d'une part, les agricultrices et, d'autre part, les actrices économiques des autres secteurs d'activité qui bénéficient aujourd'hui de ces solutions ? L'histoire nous permet d'affirmer que ce serait la meilleure façon d'assurer la relève dans ce monde agricole.

à parité pour les enfants qui relèvent du régime agricole, en finançant des initiatives locales, en construisant avec les territoires qui en sont dépourvus, en accompagnant l'expérimentation de microcrèches et en suscitant l'innovation. La MSA soutient l'ensemble des formules d'accueil des jeunes enfants en visant la réduction des inégalités territoriales et l'effectivité du libre choix des parents. La mise en place d'un congé maternité harmonisé était l'un des engagements de campagne du Président de la République. Nous avons décidé qu'il fallait en priorité s'occuper de celui des femmes

préjugé et invisibilité. Ainsi, le monde agricole n'échappe pas à ce que vivent les femmes en général, quel que soit le secteur d'activité concerné. Une fois de plus, les travaux de la délégation démontrent l'apport indéniable des femmes dans l'agriculture, comme dans tous les domaines.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour que la parité y soit respectée ? Par parité, madame la secrétaire d'État, j'entends 50 %. Ma deuxième question sera axée sur le statut juridique de la femme conjointe ou collaboratrice d'agriculteur, car beaucoup d'entre elles travaillent encore sans un véritable statut. Quelles sont vos intentions pour améliorer cette situation ? Enfin, pour présenter ma dernière question, je m'appuierai sur le témoignage

faibles revenus, retraites insignifiantes, non-reconnaissance du travail de ces femmes ... Quelles mesures comptez-vous prendre, madame la secrétaire d'État, pour apporter un peu d'espoir aux femmes agricultrices en améliorant profondément leurs conditions de vie ? J'ai entendu que vous réfléchissiez, que vous aviez travaillé sur cette question. Au-delà des réflexions, il y a

si vous me permettez cette expression, la parité est en train d'être atteinte : sur les 25 administrateurs élus, 12 sont des femmes Mais j'observe là encore la persistance de ce que l'on appelle le plafond de verre, puisque, malgré cette relativement forte proportion de femmes, le président et le vice-président sont des hommes. Pour les prochaines élections de la MSA, qui auront lieu en 2020, une réflexion est actuellement menée pour déterminer les conditions dans lesquelles pourront être appliquées les dispositions de l'ordonnance n° 2015-950 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des mutuelles. ce qui concerne les chambres d'agriculture, lors des échanges avec les syndicats dans le cadre de la préparation du prochain renouvellement des membres, le ministre de l'agriculture a proposé que les bureaux des chambres puissent appliquer la règle de mixité d'ores et déjà retenue pour l'élection des membres de chambre lors du scrutin de 2013, à savoir un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats. Tous les syndicats ont fait part de leurs difficultés. Toutefois, il nous reste encore un peu de temps pour les convaincre du bien-fondé d'une telle demande de parité dans ces instances. La parole

en 2017, 58 % seulement des agricultrices ont exercé leur droit au congé de maternité. Elles demeurent pourtant exposées à des conditions de travail difficiles, qu'il s'agisse du port de charges lourdes ou du risque d'exposition aux pesticides et aux maladies touchant les animaux. Cette situation, qui soulève de graves enjeux de santé publique pour la mère et l'enfant, s'explique par les défaillances des services de remplacement. En cas de grossesse, les employés de ces services permettent en théorie à l'agricultrice d'être remplacée dans son exploitation. Toutefois, agricultrices et syndicats agricoles ont mis en exergue l'inadéquation, voire la carence, de l'offre de remplacement, le manque d'information et les réticences psychologiques des agricultrices à laisser leur exploitation à un tiers.

les agricultrices seraient les premières à bénéficier de la mise en place du congé de maternité unique et de l'octroi d'une indemnité journalière harmonisée, quel que soit leur statut professionnel. Le monde agricole s'interroge sur la pertinence d'une telle indemnité au vu des spécificités de la profession. En effet, alors qu'un remplacement agricole coûte 145 euros par jour, les indemnités de maternité ne s'élèvent, pour les salariés du privé et du public, qu'à 80 euros

Madame la sénatrice, je rappelle que le congé de maternité de toutes les non-salariées agricoles, chefs d'exploitation, mais aussi collaboratrices ou aides familiales actuelle, la prise en charge financière par la MSA du coût du service de remplacement. J'ajoute que l'allocation de remplacement, particulièrement bien adaptée, d'après ce que nous disent les agricultrices, à l'activité agricole, n'a pas d'équivalent dans les autres régimes des indépendants ni pour aucune profession libérale. Même si le nombre de bénéficiaires a progressé de façon importante depuis 2010- 60 % de femmes ont bénéficié d'une allocation de remplacement de maternité en 2015 -, il nous faut lever tous les freins au recours au service de remplacement. Vous l'avez dit, en tant que secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, je porte le projet du Président de la République de création d'un congé de maternité harmonisé pour toutes les femmes, quel que soit leur secteur d'activité, l'idée étant de protéger les femmes et non pas les statuts. Toutes les améliorations qui peuvent être apportées pour la protection de ces femmes et de leurs enfants sont bienvenues. Je reconnais pour ma part la particularité du secteur agricole, dont les métiers justifient le maintien du recours au service de remplacement dans le cadre de la maternité. Il n'a jamais été question de le remettre en cause. Je sais que les femmes agricultrices y sont très attachées.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la délégation, mes chers collègues, mon intervention portera sur l'installation des agricultrices, et plus précisément sur leur accès aux aides à l'installation et aux terres. L'installation est un enjeu majeur pour l'agriculture dans son ensemble, alors que le nombre d'agriculteurs en Europe baisse de 25 % tous les dix ans. Les personnes qui souhaitent s'installer en tant qu'exploitante ou exploitant se heurtent à deux difficultés : d'une part, l'accès aux capitaux pour les aider à financer leurs investissements de départ et, d'autre part, l'accès à la terre, dans un contexte d'accroissement de la pression foncière. Nous avons pu le constater au travers de nos échanges avec les agricultrices, ces difficultés sont plus prononcées pour les femmes. En effet, celles qui souhaitent s'installer ne sont pas toujours éligibles aux aides à l'installation, ou le sont plus difficilement que les hommes. En 2010, seulement 28 % des nouvelles installées ont bénéficié de la DJA,

Depuis lors, les conditions d'activité minimale d'assujettissement prennent en compte des critères de temps de travail et de revenus générés en plus de la surface minimale. Toutefois, nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour juger de leurs éventuels effets bénéfiques pour les agricultrices. Mais bien souvent, les surfaces exploitées par les femmes sont inférieures à celles qui le sont par les hommes. Ensuite, le critère d'un l'âge limite fixé à quarante ans pour prétendre à cette aide peut pénaliser les femmes, dont les projets d'installation sont souvent plus tardifs que ceux des hommes. Pour prendre en compte ces spécificités, conformément aux recommandations du rapport, nous avons proposé de mettre à l'étude une évolution des critères d'attribution de la DJA, de façon à les rendre plus compatibles avec le profil des agricultrices. Nous avons ainsi proposé trois dispositions dispositions : la modulation du critère de surface d'exploitation pour l'obtention de la DJA ; le remplacement du critère d'âge limite par un critère fondé sur la notion de première installation à titre principal ; la possibilité de considérer la grossesse comme une circonstance exceptionnelle justifiant la non-réalisation

Madame la sénatrice, vous souhaitez connaître mon avis sur trois propositions relatives à l'aide à l'installation des agricultrices. La première de ces propositions concerne la modulation du critère de surface minimale d'exploitation pour l'obtention de la DJA. Vous le savez, il n'y a plus de surface minimale pour l'obtention de cette aide. Désormais, ce sont les notions de viabilité, de soutenabilité et de pérennité qui sont appréciées pour l'accès aux aides aux aides à l'installation. En effet, quelle que soit la surface de l'exploitation, il convient de permettre à un futur chef d'exploitation de vivre de son métier et de concilier ses besoins professionnels et personnels. Une exploitation de petite taille en termes de surface peut s'avérer viable en fonction des activités mises en place et des modes de production. S'agissant du critère d'âge limite, il est fixé, vous l'avez rappelé, à quarante ans par la réglementation européenne. Effectivement, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 définit un jeune agriculteur comme une personne qui n'est pas âgée de plus de quarante ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation. Une évolution de ce critère d'âge nécessite d'être abordée à l'échelle de l'Union européenne, par exemple à la faveur des discussions relatives à la PAC post-2020. Enfin, concernant la possibilité de considérer la grossesse comme une circonstance exceptionnelle justifiant le report des engagements du plan d'entreprise, sachez que la circonstance exceptionnelle ne peut être retenue que si la situation rencontrée par le jeune agriculteur répond aux conditions cumulatives suivantes ne pas être prévisible, ne pas dépendre d'une raison de convenance du jeune agriculteur et avoir des conséquences directes sur le non-respect d'un engagement. Cependant, des réflexions peuvent être menées, afin de tenir compte de l'évolution de la structure familiale pendant la période d'engagement et d'évolutions et d'évolutions majeures comme la féminisation du métier de chef d'exploitation. Une nouvelle fois, l'ouverture des échanges relatifs à la PAC post-2020 me semble être le cadre approprié pour aborder ce sujet au niveau de l'Union européenne. La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour le groupe Les Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la délégation, mes chers collègues, ma question concerne les retraites des agricultrices, en particulier des conjointes collaboratrices d'agriculteurs. de retraite figurant parmi les plus basses de toutes les catégories socioprofessionnelles. En juillet dernier, nos collègues Annick Billon, Corinne Bouchoux, Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Didier Mandelli et Marie-Pierre Monier signaient un rapport excellent, mais alarmant sur cet état de fait. Ils formulaient une quarantaine de recommandations pour sécuriser les parcours et les statuts de ces femmes, en particulier leurs retraites. En 2018, les retraites agricoles sont deux fois et demie plus faibles que la moyenne des retraites. Les retraites des agricultrices, mes chers collègues, sont souvent encore plus basses, en particulier lorsque ces femmes sont seules ou lorsqu'elles ont le statut de conjointe ou d'aide familiale. Avec environ 500 euros par mois, contre 800 euros en moyenne pour les agriculteurs, il est impossible pour ces femmes de vivre décemment. Cette différence s'explique notamment par des carrières plus courtes, un plus grand nombre d'emplois occupés et un faible niveau de cotisation. Au XXI siècle, nous ne pouvons accepter cette misère humaine et devons agir rapidement en faveur de ces femmes. Plusieurs options sont aujourd'hui sur la table des négociations une revalorisation des retraites agricoles, une évolution de leur base de calcul, le passage à une bonification forfaitaire pour enfant et une information systématique des agricultrices sur leurs statuts et leurs droits.

L'un des leviers à notre portée, c'est de combattre les inégalités persistantes en pérennisant la place des femmes dans les exploitations agricoles. Les femmes ont le choix entre trois types de statut professionnel

ni la retraite ni les accidents du travail. Une catégorie échappe à tout classement, celle des 5 000 agricultrices sans aucun statut, assumant moult responsabilités dans l'exploitation, mais très précarisées, souvent dans un grand dénuement, que l'on découvre, hélas, à l'occasion d'un veuvage ou d'un divorce. Pour pallier cette situation, la délégation propose d'engager trois types de mesures : recenser les agricultrices sans statut et déterminer avec elles celui qui leur serait le plus approprié ; sensibiliser les femmes aux préjudices sociaux qu'elles subissent par cette absence de statut ; enfin, face aux insuffisances du statut de conjoint collaborateur, la délégation préconise de le rendre transitoire pour cinq ans maximum, le temps pour l'intéressée d'affiner son projet professionnel et de choisir le statut le plus adapté à sa situation.

Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur le statut des femmes dans l'agriculture. En 1999, la création du statut de collaborateur-collaboratrice a permis d'améliorer les droits à la retraite de base,

En 2014, le plan de revalorisation a bénéficié aux collaboratrices d'exploitation en leur donnant des points gratuits de retraite complémentaire obligatoire. Pour autant, les retraites des femmes restent inférieures à celles des hommes,

remis. C'est un sujet de préoccupation pour le Gouvernement. Nous étudierons avec le ministre de l'agriculture la possibilité de travailler à un recensement. C'est pour cette raison que le Gouvernement est favorable à la limitation dans le temps du statut de collaboratrice, voire

Soulignons aussi que, si chef d'exploitation se conjugue au féminin, les capacités d'une femme et d'un homme divergent. Il est plus complexe pour une femme que pour un homme d'exercer certaines tâches très physiques. Souvent, Souvent, l'âge avançant ou bien à la suite de postures inappropriées, les agricultrices ou agriculteurs se trouvent confrontés à des complications physiques qui peuvent les empêcher partiellement d'exercer leur activité. Dès lors que le handicap touche le conjoint, c'est l'exploitante qui doit accomplir certaines tâches, avec parfois de nouvelles charges insupportables physiquement. La première des difficultés tient à ce statut de travailleur handicapé à temps partiel, qui n'existe pas dans les textes : seul un taux de handicap, variable, est reconnu, ce qui rend d'autant plus complexe l'étude des dossiers.

et de compréhension très approfondis et pertinents. Parmi les constats dressés, on relève la difficulté à concilier vie familiale et vie professionnelle. Comment en effet conjuguer une vie très prenante d'agricultrice avec un rôle tout aussi prenant de mère de famille ? Promouvoir l'attractivité du métier d'agricultrice implique, entre autres, de se poser la question de la garde d'enfants. Agriculture et ruralité vont de pair. Nous savons pourtant que les secteurs ruraux sont, en France, les plus dépourvus en termes d'outils d'accueil de la petite enfance. il a été annoncé que la prochaine convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et les caisses d'allocations familiales comportera la création de places en crèche. Celles-ci devront répondre territorialement aux besoins des parents, en lien avec les communes ou les intercommunalités. Dans le cadre de cette négociation, n'y a-t-il pas une attention particulière à avoir en matière d'accès au service public de la petite enfance, en développant de telles structures dans les secteurs ruraux ? À titre d'exemple, il conviendrait de prendre en compte les horaires de travail atypiques du secteur de l'élevage. La même problématique peut être soulevée pour l'accueil des enfants de six à dix-sept ans pour ce qui concerne l'offre de loisirs sans hébergement. Là encore, le rôle de l'État la CAF peut être décisif. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de nous donner les orientations du Gouvernement sur ce sujet.

Elles sont particulièrement adaptées aux besoins des territoires ruraux et offrent près de 2 500 places à 7 500 familles bénéficiaires. Ensuite, les LAEP, les lieux d'accueil enfants-parents, situés dans des zones rurales, sont ouverts aux enfants de moins de six ans lorsque ces derniers sont accompagnés d'un adulte, pour participer à des temps conviviaux de jeux et d'échanges. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un mode d'accueil, c'est un mode de socialisation pour les jeunes enfants et, parfois, pour les parents. les parents. Les solutions innovantes concernent majoritairement les horaires atypiques, l'accueil d'urgence, l'accueil saisonnier, les horaires extrêmes, l'accueil les week-ends et les jours fériés et l'accueil des enfants différents en milieu ordinaire. Depuis 2016, une centaine d'innovations ont ainsi été repérées et répertoriées. En partageant l'expérience acquise et grâce à un nouveau dispositif, la MSA veut favoriser l'émergence de nouveaux projets, qui participeront à la qualité de vie des familles dans les territoires ruraux. Plus récemment, elle a contribué à la mise en place de haltes-garderies itinérantes, qui sont hébergées dans des bus circulant de commune en commune. Vous m'interrogez

La MSA apporte un soutien financier à quelque 30 000 familles, pour environ 4,5 millions d'euros en 2016. La très grande majorité des ALSH en zone rurale accueille sans distinction les enfants de trois à onze ans, et la moitié propose des activités au-delà de onze ans.

Vous me pardonnerez de m'éloigner légèrement des quarante préconisations pour aborder un autre sujet, celui des femmes et de l'agriculture biologique, que le rapport évoque sans l'approfondir, faute de données suffisantes. Néanmoins, le dernier recensement agricole de 2010, mentionné dans ce document, révèle que, parmi les exploitations agricoles gérées par des personnes de moins

Les pistes d'explication pour décrire ce phénomène sont balbutiantes, et la Fédération nationale d'agriculture biologique enquête actuellement sur ce sujet. Les résultats de ce travail seront présentés à l'occasion d'un colloque le 10 avril prochain. Aussi, pour éviter de tomber dans le stéréotype de genre, nous nous concentrerons sur les facteurs socio-économiques, plus objectifs. 30 % à 50 % des agriculteurs et agricultrices bio se lancent hors cadre familial. Nous connaissons tous le problème de l'accès au foncier. Il est bien plus aisé, pour commencer, d'acquérir une petite parcelle plutôt qu'une exploitation importante. Or, sur de petites surfaces, le bio, associé aux circuits courts, est bien plus rentable que le conventionnel. L'agriculture bio est également nettement moins mécanisée, ce qui nécessite un apport en capital moindre. L'activité est plus facilement diversifiable- agrotourisme, vente directe On le voit, sans même prendre en compte d'autres considérations telles que la santé, le respect de la terre ou la qualité des produits, il est moins coûteux de se lancer en bio. Cet intérêt économique se traduit manifestement par un bien meilleur accès des femmes au statut d'exploitante.

bio et lutte contre les stéréotypes de genre, si l'on peut le formuler de cette manière. Vous avez raison, les femmes s'engagent tout particulièrement dans l'agriculture biologique. D'ailleurs, les exploitations agricoles que j'ai eu l'occasion de visiter depuis que je suis en

protections est souhaitable pour les femmes comme pour les hommes dans les exploitations agricoles. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la délégation, mes chers collègues, alors que le nombre d'agriculteurs diminue de 25 % tous les dix ans en Europe, il est impératif de favoriser l'insertion de nouveaux exploitants, en particulier celle des femmes. Les agricultrices se heurtent à des difficultés d'installation plus prononcées que celles que rencontrent leurs homologues masculins, car elles héritent rarement d'une exploitation et font face à des coûts d'accès à la terre et aux capitaux très élevés. Afin de lutter contre ces inégalités, des dispositifs d'aide ont été mis en place, comme la dotation jeunes agriculteurs, la DJA, qui garantit un soutien financier en cas de première installation. Dans les faits, une partie des agricultrices se trouve cependant exclue de l'accès à cette dotation, en raison de critères d'attribution rigides et inadaptés. Pour en bénéficier, il faut en effet exploiter une surface minimale,

les possibles maternités, qui peuvent retarder l'âge de l'installation et la mise en oeuvre du plan. À l'aune de ces incohérences, la délégation aux droits des femmes préconise d'adapter les conditions d'attribution de la DJA au profil des agricultrices, en aménageant le plan d'entreprise en cas de grossesse, ou en remplaçant le critère d'âge limite par un critère fondé sur la notion de première installation à titre principal. Madame la secrétaire d'État, quelles mesures envisagez-vous de prendre afin de faciliter l'installation des agricultrices ? La parole est

mais aussi dans l'aspect très, n'ayons pas peur des mots, dudit projet. Les bonnes pratiques et les capacités d'innovation pédagogique de l'enseignement agricole en matière d'éducation à l'égalité entre

Un exemple : le colloque mené au lycée viticole de Mâcon, avec des témoignages forts, posant la question des préjugés sur les stéréotypes de genre et la manière dont on peut mieux accompagner les jeunes filles dans la création ou la reprise

en particulier d'avoir ouvert à la réflexion du point de vue féministe des champs quasiment en jachère jusqu'ici. Parmi toutes les recommandations formulées par la délégation, je retiens la trentième, celle qui a trait à la santé des femmes agricultrices. Le rapport préconise la mise en oeuvre d'une évaluation scientifique des conséquences, sur la santé maternelle et infantile, et plus généralement sur l'organisme des femmes, de de l'exposition aux produits utilisés : manipulation de médicaments vétérinaires, utilisation de pesticides- vous venez d'évoquer la question, madame la secrétaire d'État. La Haute Assemblée a très récemment débattu de la proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes de produits phytopharamaceutiques. Ces échanges nous ont permis de mesurer pleinement les responsabilités des autorités, du monde agricole et des industriels en matière de prévention sanitaire. Si de tels dispositifs d'indemnisation peuvent être mis en place, c'est parce qu'il existe désormais une connaissance scientifique suffisamment large des phénomènes, de l'impact des molécules phytosanitaires et des précautions à prendre. Très récemment, et encore ce matin, la presse révélait les dernières avancées de la recherche française, mettant en évidence les effets toxiques de l'exposition aux pesticides. Le même effort doit être engagé pour mieux connaître les effets des médicaments vétérinaires et des produits phytosanitaires sur les femmes agricultrices enceintes, sur le développement de leur foetus, voire sur les difficultés- certaines personnes ont témoigné en ce sens

du débat. Vous avez raison de le souligner, c'est la connaissance scientifique qui nous a permis de disposer d'une appréhension vraiment fine des conséquences de l'utilisation de ces produits et de mettre en place un système de protection des femmes contre les produits phytosanitaires et contre les pesticides. J'ai rappelé tout à l'heure l'existence du plan Écophyto 2+, visant, disais-je, à réduire l'utilisation de ces produits et surtout à supprimer celle des plus dangereux d'entre eux. Je veux rappeler également que le code du travail impose que les machines et les équipements de travail soient conçus de manière à ne pas exposer les utilisateurs à des risques pour leur santé et pour leur sécurité.

de grossesse et de développement de l'enfant. Les risques sont multiples, mais les connaissances scientifiques, bien qu'elles progressent considérablement, restent insuffisantes pour pouvoir les évaluer d'une manière pleinement satisfaisante

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, mes chers collègues, je salue l'initiative d'organiser un débat sur les femmes et l'agriculture. Les questions, en la matière, ne manquent pas : les petites retraites agricoles, la formation professionnelle notamment. À mon tour, mes chers collègues, je souhaite rendre hommage à toutes ces femmes agricultrices et femmes d'agriculteurs dont le courage et la force font toute mon admiration. Je sais la place qu'elles occupent dans l'agriculture française, particulièrement dans mon département, très agricole, la Mayenne. Je souhaite rendre hommage, donc, à toutes ces femmes souvent qualifiées d'« invisibles », qui travaillent dans l'élevage, la viticulture, le maraîchage et autres cultures, dans des conditions physiques et psychologiques parfois difficiles, et dont le statut n'a pas été, pendant trop longtemps, reconnu. Oui, la vie de ces femmes est faite de sacrifices et d'engagements forts, de passion. La féminisation du milieu agricole augmente. On ne peut que s'en féliciter. Deux exemples me semblent significatifs : un quart des dirigeants ou codirigeants d'exploitation agricole sont des femmes ; le nombre de femmes qui font librement le choix de devenir agricultrice ne cesse d'augmenter. Bien souvent, la question de la conciliation entre les vies professionnelle et personnelle se pose, notamment pour les femmes qui sont mères ou qui souhaitent le devenir. Cette question représente aussi un frein, pouvant éveiller la réticence de celles qui désireraient exercer cette profession.

Aujourd'hui, c'est à un risque sanitaire que nous sommes confrontés : 58 % des femmes agricultrices qui attendent un enfant ne prennent pas leur congé de maternité, parce qu'elles sont mal informées sur leurs droits, ou encore en raison du coût

L'année dernière, madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous avez annoncé la mise en place d'un projet pilote au sein du ministère de l'agriculture en matière de budget « genré

clé dans le combat pour l'égalité, en ce qu'elle permet de donner la parole aux femmes, de susciter des vocations, d'inspirer, d'illustrer des réussites au féminin. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juin 2012 et de la loi du 4 août 2014, les chambres d'agriculture

n'ont fait l'objet d'aucune obligation juridique- vous y faisiez référence tout à l'heure, madame la secrétaire d'État. À titre d'exemple, le conseil d'administration de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, l'APCA, ne compte qu'une femme pour trente-trois hommes, et son bureau, une

au sein des instances dirigeantes des différentes chambres d'agriculture, de l'APCA, des syndicats agricoles, des coopératives agricoles. Madame la secrétaire d'État, une modification de la loi est-elle envisagée sur ce plan ? mettre en oeuvre pour encourager la féminisation de la gouvernance professionnelle ? Plusieurs leviers existent : rôles modèles, réseaux féminins, meilleure répartition des tâches dans la cellule familiale pour libérer du temps libre, législation, etc. La parole est à Mme la secrétaire Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice, vous posez une question cruciale. Je ne reviens pas sur le constat, puisque vous l'avez très justement dressé. La parité complète sur les listes électorales sera atteinte à compter du deuxième renouvellement des chambres départementales d'agriculture et des chambres régionales d'agriculture qui suit la promulgation de la loi, soit en 2020- les prochaines élections des chambres d'agriculture auront lieu en 2019. la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, que j'évoquais tout à l'heure, est inscrite l'amélioration de la représentation des femmes au sein des SAFER, les sociétés

Vous conviendrez aisément qu'il en est ainsi de la politique comme de l'agriculture. Aussi ne peut-on que se féliciter de l'excellent travail effectué par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les femmes et l'agriculture ; la présentation de son rapport vient aujourd'hui clôturer un cycle de plus d'un d'un an de colloques, de rencontres, d'auditions et de témoignages, au plus près de la réalité des agricultrices et de leurs territoires. C'est donc avec fierté que la fille d'agricultrice que je suis souhaite se faire l'écho de la recommandation 34 dudit rapport, visant à encourager les jeunes filles à choisir le métier d'agricultrice. Il s'agit d'un métier certes exigeant, mais ô combien prioritaire en matière d'économie, d'écologie, et surtout de santé publique. Aussi est-il primordial de susciter des vocations et d'orienter les jeunes filles vers ces filières malheureusement peu ou mal connues,

des professionnels de l'éducation et de l'orientation sur les débouchés dans le milieu agricole ; en communiquant sur tous les supports, y compris sur internet et les réseaux sociaux, avec un vocabulaire adapté et des images s'adressant tant aux filles qu'aux garçons ; en valorisant davantage les bonnes pratiques et en insistant sur les aides à l'installation et les moyens existant pour accompagner les jeunes agricultrices et agriculteurs ; en créant, enfin, des internats et des structures d'accueil et d'hébergement adaptés aux filles, tant en formation initiale qu'en formation continue. À n'en pas douter,

Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur les actions conduites par le Gouvernement pour la diversification des choix d'orientation scolaire et professionnelle en direction des jeunes filles. Le réseau Insertion-égalité des chances anime des actions de sensibilisation spécifiques et des appels à projets auprès des établissements, pour faire réfléchir à la fois les élèves et l'ensemble du monde éducatif à ce sujet. À titre d'exemple, le projet Filagri accompagne les filles minoritaires dans leur formation ; il a mobilisé huit régions pendant quatre ans. Un guide à destination des équipes, dans les établissements, vise également à mieux accompagner les apprenants dans leurs projets personnels, scolaires et et professionnels. Il a été conçu avec une attention spécifique à l'égalité entre filles et garçons, pour encourager l'orientation des jeunes filles en direction de ces filières. Je crois, comme vous, madame la sénatrice, à l'importance des rôles modèles. C'est pour cette raison que nous renforçons notre communication destinée à valoriser des femmes qui exercent des métiers dans lesquels les hommes sont fortement représentés,

particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Enfin, le Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes a fortement mobilisé les lycées agricoles, qui ont travaillé dans ce cadre au regard porté sur les métiers de l'agriculture par les jeunes. La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, pour le groupe Les Républicains. madame la présidente de la délégation, mes chers collègues, ce rapport, dont je salue moi aussi la pertinence, nous permet de mesurer le chemin parcouru depuis les années 1960 pour faire progresser les droits et la condition des femmes agricultrices. Mais, mes chers collègues, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Le tableau qui y est peint nous appelle également à nous retrousser les manches, tant les actions à mener sont structurantes. En 1949, Simone de Beauvoir écrivait : « C'est le travail qui peut seul garantir à une femme une liberté concrète. » Cette liberté demeure à conquérir pour les femmes agricultrices. En effet, les conditions dans lesquelles celles-ci exercent leur métier nous interpellent, diront certains, nous révoltent, diront d'autres. La faiblesse des revenus a des répercussions sur leur statut, leur protection sociale et le montant de leur retraite. Si cette problématique n'est pas exclusivement féminine, elle se pose avec d'autant plus de vigueur pour les femmes agricultrices en raison de la création récente du statut de conjoint collaborateur et de l'accès tardif au statut de chef d'exploitation. Les chiffres sont éloquents : la retraite moyenne d'une femme agricultrice se situe entre 500 et 600 euros. Le minimum vieillesse, quant à lui, est d'environ 800 euros.

particulier la question des retraites. Je ne me répète pas : j'ai parlé tout à l'heure des pistes de travail sur lesquelles planche le Gouvernement, avec notamment le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. Mais j'entends bien votre interpellation et vous assure une nouvelle fois qu'il s'agit d'un sujet majeur sur lequel l'ensemble du Gouvernement est mobilisé. La parole

d'étendre le dispositif de remplacement ou de mettre en place un chèque emploi service prépayé utilisable pour la garde d'enfants, mais également

des dispositifs de remplacement, dont le coût serait pris en charge, comme pour les maternités, en cas d'enfant malade. J'ai évoqué tout à l'heure la question des bus itinérants et des modes d'accueil innovants. Actuellement, vous savez que seul le congé de maternité est pris en charge par la MSA. En cas de maladie très grave, il est possible de bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale ; ce droit est ouvert aux personnes qui assurent la charge d'un enfant gravement malade. Mais cette allocation ne permet bien sûr pas de financer le remplacement de la mère

effet, il faut se former pour s'installer tout en faisant face à une charge de travail importante et à une administration qui prend toujours plus de temps et de place ! Même s'il est souvent une passion, ce métier doit s'accompagner d'une meilleure protection sociale et d'un vrai statut. L'exploitation familiale d'autrefois

Dans la région Pays de la Loire, la démarche des agricultrices est souvent tournée vers le qualitatif et les circuits courts ; je pense notamment aux filières du sel, de l'élevage, du maraîchage ou de la viticulture. Parmi les quarante recommandations du rapport, il me semble que les points suivants sont prioritaires et demandent que des solutions soient mises en oeuvre très rapidement. d'abord, au statut, avec un parcours de formation initiale adapté. Je pense, ensuite, à la revalorisation du montant de base des retraites agricoles, incluant une bonification forfaitaire

Vous le savez, les femmes, qui représentent 30 % des contributeurs au fonds de formation, n'en bénéficient qu'à hauteur de 9 %, contre 14 % globalement. VIVEA, qui est le fonds de formation des agriculteurs, mène une action spécifique sur le sujet.

Cette constatation souvent évoquée doit rester dans nos esprits. L'épouse du chef d'exploitation a longtemps été considérée comme sans profession.

Aujourd'hui, elles souhaitent un véritable statut qui leur assure une protection sociale adaptée et une retraite calculée sur les meilleures années de leur vie professionnelle. Afin de survivre à l'agriculture, l'équilibre se fait souvent par l'exercice d'un métier extérieur. Je salue le mérite de ces femmes qui composent ainsi entre deux mondes, permettant très souvent de sauver l'exploitation. Un couple d'agriculteurs vit en moyenne, selon une récente enquête de la MSA effectuée en 2017, avec à peine 354 euros par mois. Telle est la vérité, madame la secrétaire d'État ! Dès lors, comment valoriser la féminisation croissante de la profession agricole et encourager l'accès des femmes aux responsabilités dans les instances agricoles ? Cette démarche est indispensable. Les femmes apparaissent comme les nouveaux catalyseurs du monde agricole. Je considère que leur avenir dépend d'une solide formation. Elles pourront davantage reconvertir une partie du secteur agricole en secteur de services. Favoriser leur installation permettrait de pérenniser les exploitations, sans négliger pour autant la production. Pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, nous indiquer le plan envisagé par le Gouvernement pour conforter la place des exploitantes agricoles, qui, de jour en jour, font vivre le tissu rural ? ? Quelles sont les suites proposées pour les aides à l'entrepreneuriat ou le remplacement en cas de congé de maternité et l'aide à domicile ? Enfin, quelles mesures d'action locale adaptées à chaque territoire rural proposez-vous ? La parole est à Mme la secrétaire

très concret, elles sont l'ADN même de cet enseignement agricole. Elles cherchent à développer l'autonomie des jeunes femmes, à les rendre actrices de leur parcours, de leur formation et, plus généralement, de leur parcours professionnel. Tel me paraît vraiment être le fil rouge de tous les sujets que vous évoquez, monsieur le sénateur : l'autonomisation, l'émancipation

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer à mon tour l'excellent travail réalisé par nos collègues de la délégation aux droits des femmes. Le thème des femmes et de l'agriculture, qui a donné lieu l'an dernier à un colloque et à un rapport d'information, permet de mettre un éclairage sur une réalité mal connue et sur des situations qu'il convient de corriger. C'est pourquoi j'espère que de nombreuses préconisations qui ont été formulées et qui relèvent, pour bon nombre d'entre elles, du bon sens paysan, seront retenues. On ne peut que se réjouir, en effet, du nombre de femmes qui rejoignent chaque année le monde agricole en France. Elles entendent mener un projet professionnel qui est aussi le choix d'un mode de vie et qui a été très souvent mûrement réfléchi. Les femmes s'installent souvent plus tard que les hommes et avec un niveau d'études supérieur. Autrement dit, à l'issue d'un cursus plus complet, les nouvelles agricultrices ont une formation qui leur permet de mettre en place des projets innovants, lesquels s'inscrivent davantage dans l'air du temps et répondent mieux aux attentes des consommateurs. C'est ainsi que, en 2017, dans mon département, les Hautes-Alpes, sur 47 nouvelles installations, 17 ont des femmes comme chef d'exploitation. Le pastoralisme n'est pas en reste puisque de plus en plus de jeunes femmes se destinent au métier de bergère ou d'aide-bergère. Cette proportion peut même atteindre les deux tiers selon les territoires. Or le plan Loup 2018-2023 vient de mettre un coup d'arrêt à cette dynamique. Aucune avancée significative n'a été réalisée pour défendre les troupeaux. Le dispositif d'utilisation du tir de défense est toujours aussi contraignant pour les éleveurs et les mesures d'effarouchement ont montré leurs limites, avec des attaques de plus en plus nombreuses, puisque 10 000 animaux ont été tués par le loup en 2017